par lettre en date de ce jour, le Gouvernement sollicite l'inscription, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire à l'ordre du jour du jeudi 14 juin matin. Nous pourrions fixer le début de l'examen de ce texte à dix heures trente, avant la suite de la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Y a-t-il des observations ? observations ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées, présentée par M. Alain Milon et plusieurs de ses collègues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

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a adopté le 30 mai dernier, à l'unanimité, la proposition de loi de notre collègue Alain Milon qui autorise les examens génétiques dans l'intérêt thérapeutique des proches des personnes décédées. L'évolution proposée s'inscrit dans le prolongement de la consécration, en 2004, d'une obligation d'information de la parentèle en cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave susceptible de mesures de prévention ou de soins. Le texte ne modifie pas le point d'équilibre alors défini par le législateur entre le secret souhaité par le patient, d'une part, et le devoir moral de solidarité familiale, d'autre part. Il tire les conséquences du caractère définitif des résultats des examens génétiques, qui ont ceci de particulier qu'ils peuvent avoir des conséquences non seulement pour la personne testée, mais aussi pour la famille. Son objectif est d'éviter les situations de perte de chance. La commission des affaires sociales est convaincue de l'avancée majeure que permettrait l'adoption de cette proposition de loi. Elle a néanmoins jugé indispensable de prévoir un dispositif rigoureusement encadré, fondé sur le respect de deux principes fondamentaux la protection de la volonté et de la dignité de la personne décédée et la garantie d'une prise en charge de qualité pour les familles. Pour atteindre cet objectif, elle a apporté deux séries de précisions. S'agissant tout d'abord des conditions dans lesquelles un examen génétique peut être réalisé sur une personne décédée dans l'intérêt médical d'un tiers, elle a défini quatre conditions cumulatives. En premier lieu, la personne décédée ne doit pas avoir, de son vivant, exprimé son opposition à cet examen. Par parallélisme des formes, nous retenons ici le même régime de consentement présumé que celui qui est prévu par la loi pour le don d'organes. En second lieu, l'examen est réalisé à des fins médicales dans l'intérêt des ascendants, descendants et collatéraux de la personne décédée. La finalité de l'examen doit, en toute circonstance, demeurer l'intérêt médical des personnes partageant un lien de sang avec la personne décédée. En troisième lieu, l'examen est réalisé à la demande d'un membre de la famille potentiellement concerné par l'identification d'une anomalie génétique chez la personne décédée. En dernier lieu, il est prescrit par un médecin qualifié en génétique ou membre d'une équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin qualifié en génétique. En tout état de cause, il reviendra au médecin prescripteur d'apprécier si les conditions sont réunies, en particulier celle relative à l'intérêt de la parentèle. En ce qui concerne les circonstances médicales dans lesquelles l'examen peut être effectué, comme l'a indiqué l'Agence de la biomédecine, deux situations doivent être distinguées. L'examen doit être possible à partir d'éléments du corps prélevés préalablement au décès de la personne. Cette situation se présentera le plus souvent en oncologie. Il convient en outre d'autoriser l'examen dans le cadre d'une autopsie médicale : je pense ici notamment aux cas de mort subite chez des sujets jeunes, qui peuvent résulter d'une pathologie cardiaque susceptible de concerner également la fratrie. Le cas échéant, la famille de la personne décédée, en particulier ses frères et soeurs, pourrait être orientée vers un conseil génétique. La proposition de loi adoptée par la commission des affaires sociales est fortement attendue par les professionnels de santé, tous soucieux d'améliorer les prises en charge. L'Agence de la biomédecine y voit une évolution fondamentale de notre droit. À mon sens, ce texte est en effet l'une des contributions que nous pouvons apporter au renforcement de la politique de prévention dans notre pays. Je sais, madame la ministre, que l'investissement dans la prévention, qui demeure le parent pauvre de notre système de santé, est l'une de vos priorités. Le dispositif proposé est également attendu par les professionnels, parce qu'il apporte une clarification bienvenue. Il semble en effet que les pratiques médicales se caractérisent par une certaine hétérogénéité, ce qui est source à la fois d'inégalités et de pertes de chance. Enfin, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, parmi les nombreuses questions soulevées en génétique dans la prochaine révision des lois de bioéthique, cette proposition de loi concerne un sujet bien circonscrit. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un dispositif consensuel et fortement attendu. Les conditions sont donc réunies pour avancer sans attendre. Il serait dommageable que de simples considérations de forme ou de calendrier nous fassent courir le risque de retarder des prises en charge qui pourraient s'avérer nécessaires.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les évolutions et la mise au jour de techniques nouvelles dans le domaine de la génétique soulèvent des questions inédites qui interpellent à juste titre le législateur. Nos débats ont une résonance particulière, alors que le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, m'a remis hier le rapport de synthèse des états généraux de la bioéthique. Leurs travaux, qui ont débuté au mois de janvier, ont associé des citoyens, des associations, des sociétés savantes de professionnels de santé, des scientifiques et différents courants de pensée afin de recueillir un large panorama d'opinions de la société et, surtout, de répondre à la question : « Quel monde voulons-nous pour demain ? » La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui tend, pour sa part, à répondre à un problème très précis, puisqu'il s'agit d'autoriser la réalisation d'examens de génétique après le décès d'une personne- ce que les lois de bioéthique, et en particulier les dispositions qui encadrent le consentement à la réalisation d'un examen de génétique, ne permettent pas aujourd'hui. Je comprends bien votre démarche, dictée par le souci de prévenir d'éventuels risques et d'accompagner l'évolution technique. Les progrès de la génétique- et nous pouvons nous en réjouir -permettent, en effet, de plus en plus d'analyser les caractères héréditaires prédisposant à la survenue de certaines pathologies, notamment des cancers. Toutefois, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer en commission, je regrette que le débat sur ces sujets de bioéthique débute au Sénat sur cette question précise, alors même que plusieurs rapports sont encore attendus. Je pense, en premier lieu, à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, qui sera rendu à la fin de l'été, mais également au rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPECST, et au rapport du Conseil d'État. Je reste certaine que le vecteur le plus approprié pour la réforme que vous envisagez est la loi de bioéthique, dont les travaux parlementaires devraient commencer d'ici quelques mois. mois. À échéances définies, il est ainsi prévu que les lois de bioéthique soient revues afin d'assurer la meilleure adaptation entre l'éthique et le progrès technique. À ce titre, ce sont ces lois qui garantissent la prise en compte de l'ensemble des implications des questions très sensibles et très complexes que vous soulevez. Vous abordez par exemple, à l'article 2 de la proposition de loi, les modalités de conservation des échantillons après le décès d'une personne et vous confiez à l'Agence de la biomédecine l'édiction de règles de bonnes pratiques. en parallèle, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique sur cette question précise de la durée de conservation des échantillons biologiques. Le sujet n'est pas simplement technique : il touche au consentement en génétique et à l'information des membres de la famille en cas d'anomalie génétique, qui sont au coeur même de l'édifice bioéthique. Une modification de ce cadre comme de celui de l'information de la parentèle ne peut être traitée de façon isolée, c'est-à-dire sans prendre en compte l'ensemble des problématiques dans le domaine de la génétique, dans le contexte de la médecine génomique, prédictive en l'occurrence. Je suis favorable au principe d'ouvrir la possibilité, de façon encadrée, de réaliser des examens de génétique, alors que la personne est décédée, mais il me semble qu'il convient d'en débattre dans le cadre prévu à cette fin, à savoir la révision de la loi de bioéthique, en ayant une vision de l'ensemble des enjeux et impacts. Le débat est de toute façon ouvert et je suis sûre que vos réflexions pourront nourrir le projet de loi dès qu'il sera déposé au Parlement. La parole

Les nombreuses auditions menées confirment toutes la forte attente des professionnels de santé, qui y voient une avancée majeure. L'évolution législative permettra une harmonisation des pratiques et donc une plus grande égalité entre les patients. Notre capital génétique peut nous prédisposer en effet au développement de certaines maladies potentiellement graves, voire mortelles. C'est le cas par exemple de certaines formes de cancer du sein. Connaître l'histoire génétique ou le génome d'une tumeur revêt plusieurs avantages pour le patient, mais également pour sa famille. Dans certains cas, cela permet de mieux cibler le traitement et d'augmenter les chances de guérison. C'est tout l'enjeu actuel des nouvelles thérapeutiques qui révolutionnent la prise en charge et le pronostic de certains cancers. Connaître l'histoire génétique peut être également nécessaire dans certaines situations, dans le cas de maladies à forte présomption héréditaire, afin de remonter l'histoire familiale de cancers pour dépister plus précocement la maladie chez les apparentés vivants, mieux les informer et proposer des mesures de prévention. Jusqu'à présent, la loi prévoyait que ces tests génétiques ne pouvaient être réalisés que dans l'intérêt de la personne malade. La notion d'obligation d'information de la parentèle en cas de maladie génétique grave susceptible de mesures préventives ou thérapeutiques, dans le respect du droit du patient à ne pas être informé lui-même, est apparue dès 2004. Tout en conservant cet équilibre, la proposition de loi permet la réalisation d'un examen génétique sur une personne décédée, au bénéfice des membres de la famille. Cet examen, jusqu'ici impossible, entraîne des pertes de chance pour certains patients susceptibles de bénéficier d'un diagnostic précoce. Nous devons remédier à cela. C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi, dont la rédaction initiale pouvait laisser planer quelques doutes quant aux conditions de réalisation des examens et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être demandés. Les amendements votés en commission permettent de préserver les grands principes éthiques. Concernant le respect de sa volonté, sur le même modèle que le don d'organes, le patient pourra signifier son opposition à un examen génétique de ses tissus. Si aucune opposition n'a été formulée, l'examen pourra alors être réalisé après son décès, uniquement à des fins médicales et dans l'intérêt des personnes liées à lui par le sang. Si l'examen peut être demandé par un membre de la famille potentiellement concerné, seul un médecin qualifié en génétique ou un collège de médecins comprenant au moins un généticien peut le prescrire. Il est important de le préciser, l'examen se fera nécessairement sur des tissus prélevés avant le décès ou lors d'une autopsie, pour les cas de mort subite notamment chez les sujets jeunes. J'ai entendu la position du Gouvernement, qui nous propose d'inscrire cette mesure dans le cadre de la loi sur la bioéthique, laquelle sera présentée au Parlement en 2019.

une perte de chance pour bon nombre de nos concitoyens, car un délai de plusieurs mois peut mettre en jeu un pronostic vital. Cette proposition consensuelle, attendue, qui a recueilli l'unanimité en commission, pourrait être appliquée sans délai grâce à ce texte.

les conclusions des états généraux de la bioéthique organisés par le CCNE, nous voici réunis pour débattre d'un sujet qui concerne, lui aussi, les problématiques de génétique et de génomique. En effet, la proposition de loi relative à l'autorisation des examens des caractéristiques génétiques sur les personnes décédées de M. Milon et de ses collègues, rapportée par Mme Deroche, s'inscrit au coeur de la bioéthique. On pourrait douter de l'opportunité d'étudier un tel texte en dehors des débats qui se tiendront lors de la révision des lois de bioéthique à venir, débats que je souhaite le plus apaisés possible. ! je crains que les passions ne prennent le pas sur la raison- cela peut arriver, madame la ministre -et j'accueille donc favorablement l'étude de telles dispositions dès aujourd'hui. Ce qui est fait est fait Les éléments contenus dans le texte relèvent d'un ajustement presque technique de la législation actuelle. Comme vous le savez, les progrès en génétique et en génomique des dernières années sont considérables. Imaginez-vous que moins de cinquante ans séparent la découverte du caryotype humain, en 1956, du premier séquençage complet de l'ADN du génome humain, en 2003 Comment croire que, il y a à peine vingt ans, les premiers cancers d'influence génétique étaient mis au jour, les premières controverses apparaissant également- sur la brevetabilité du vivant, notamment ? Depuis lors, les politiques de santé publique ont été adaptées et ont pris en charge les personnes ayant un risque accru de développer certains cancers ou d'autres pathologies. Grâce à la connaissance d'un facteur de risque- ici génétique le suivi est adapté, voire personnalisé, et l'équipe médicale pourra prendre des mesures de prévention ou effectuer des soins spécifiques qui influenceront grandement le pronostic du patient. Il s'agit non pas simplement d'identifier la présence ou non d'une mutation pathologique d'un gène, mais d'expliquer les conséquences de cette présence, les risques induits et la prise en charge qui en découlera. Le simple résultat ne saurait être appréhendé par la personne seule. La présente proposition de loi cherche à permettre la réalisation de certains tests génétiques sur une personne décédée dans « l'intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux ». Cette proposition équilibrée respecte toutefois la volonté du patient qui se serait exprimée de son vivant contre la réalisation de tels tests. une fois de plus, dans sa grande sagesse, s'honore en répondant à une attente des professionnels pour une meilleure prévention. Il faudra que le législateur demeure vigilant sur ces questions d'utilisation de tests génétiques, leur nombre et leur finalité, car la baisse de leur coût et leur disponibilité en libre accès dans certains pays ne doivent pas laisser penser que l'information brute d'un résultat puisse être bien appréhendée par tout un chacun. En plus de s'interroger sur la protection de données aussi personnelles que l'identification génétique, il convient de continuer à réserver la réalisation de tels tests au sein d'un dispositif médical de consultation génétique, de préférence pluridisciplinaire. chers collègues, ce texte relève bien évidemment de la bioéthique et représente une avancée qui aurait le mérite d'être adoptée en dehors de tout débat trop passionné. Il étend, mais de manière stricte, une technique existante, prévue dans un parcours précis, encadrée par des professionnels de santé en demande de ces outils.

de loi déposée par le président Alain Milon et plusieurs de ses collègues a un caractère extrêmement important, avec des enjeux essentiels en termes de santé publique et de bioéthique. Comme l'a très bien expliqué la rapporteur, Catherine Deroche, l'objectif de cette proposition de loi est de répondre à un manque législatif, qui fait qu'actuellement le consentement d'un patient doit être clairement exprimé pour mener sur sa personne des examens de caractéristiques génétiques. Bien évidemment, ce consentement est impossible à obtenir une fois la personne décédée. Lever cette limite et instaurer un régime de consentement présumé va donc permettre de transmettre des informations médicales cruciales aux membres de la famille potentiellement concernées par des maladies génétiques, des maladies héréditaires. On sait d'emblée combien ce genre de sujet peut être sensible, car touchant à l'intime. Il aurait pu effectivement, comme l'aurait sans doute préféré Mme la ministre, être abordé lors de la révision des lois de bioéthique d'ici quelques mois. mois. Il est donc important que nous rassurions ici nos concitoyennes et nos concitoyens : il n'est nullement question d'atteinte à la dignité et à l'intégrité humaines. Ces analyses, réalisées à des fins purement médicales, sont bel et bien faites dans le respect des protocoles fixés par l'Agence de la biomédecine, dans l'intérêt des descendantes et des descendants, des proches, dans un souci de prévention, de surveillance. Comme cela est précisé dans le rapport de notre collègue, les analyses sont donc faites dans deux cadres très précis : soit à partir d'éléments du corps prélevés préalablement au décès de la personne- dans ce cas, la personne a fait l'objet d'un prélèvement tissulaire ayant conduit au diagnostic le prélèvement a été conservé par le laboratoire ; la personne est ensuite décédée et le médecin qualifié en génétique prescrit, dans l'intérêt de la parentèle, l'examen des caractéristiques génétiques de la personne décédée à partir du prélèvement conservé - ; soit dans le cadre d'une autopsie médicale- le prélèvement est alors quasi concomitant au constat de décès ; cette possibilité vise principalement les situations de mort subite, en particulier des sujets jeunes. Mais le texte, dans sa version originelle, pouvait induire, voire entraîner des dérives. Aussi, je salue le travail de réécriture mené par notre rapporteur Catherine Deroche, qui permet de le clarifier, dans le respect des droits de la personne. En effet, toute personne peut, de son vivant, signifier son refus que de telles analyses soient effectuées une fois qu'elle sera décédée. Cela est également vrai pour la levée du secret médical : la personne peut s'y opposer. Cela permet ainsi de garantir les libertés individuelles, ce qui est primordial en ce domaine. Le texte issu des travaux de la commission permet également de ménager un équilibre entre la possibilité du secret et le droit pour la famille de savoir. Les progrès médicaux et scientifiques en génétique sont tels aujourd'hui qu'il serait dommageable de ne pas faire évoluer notre loi afin de développer la prévention. Plus de 6 000 maladies génétiques sont aujourd'hui répertoriées et le champ des connaissances n'en sera que plus large et meilleur avec les nouvelles possibilités offertes par le cadre J'en profite, madame la ministre, pour souhaiter que, conformément à vos engagements, des actes forts soient posés par le Gouvernement pour dégager des moyens humains et financiers afin de développer, au coeur de notre politique de santé, la prévention. En résumé, le groupe CRCE se prononcera favorablement sur cette proposition de loi, qui, je l'espère, ira jusqu'au bout de son parcours législatif pour permettre une meilleure prise en charge médicale de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales,

Au lendemain de la présentation du rapport des états généraux de la bioéthique, qui se sont tenus de janvier à mai, nous sentons bien que ces sujets sont au coeur de l'actualité. Un grand quotidien national en a fait d'ailleurs sa une. De nombreux clivages existent dans notre société sur des problématiques telles que la fin de vie ou l'assistance médicale à la procréation et ils sont loin d'être tranchés. Espérons, comme l'a dit notre collègue, que nous pourrons en discuter avec raison et sans trop de passion dans quelques mois. La commission des affaires sociales s'est réunie le mercredi 30 mai pour examiner la proposition de loi déposée par notre collègue Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, visant à autoriser les analyses génétiques sur personne décédée. Je ne vous cache pas, mes chers collègues, que je n'ai pas tout de suite mesuré la portée de ce texte. C'est en commission, après avoir écouté attentivement les débats, Mme la rapporteur, Mme la ministre, dont les explications ont été très claires, que j'ai compris que cette proposition de loi portait une véritable évolution.

il doit être capable d'en comprendre les changements et les mutations pour accompagner le progrès et l'encadrer. Tel est l'objet de ce texte : permettre à chacun de disposer d'une meilleure information médicale concernant une personne décédée, tout en respectant naturellement la volonté de la famille et les prescriptions médicales des médecins.

Les nombreuses évolutions scientifiques et, plus particulièrement, les avancées de la médecine changeront notre rapport au monde et au corps humain ; ce sera notre rôle de parlementaires d'accompagner ce changement. Lors de son audition au Sénat, Mme Anne Courrèges, directrice de l'Agence de la biomédecine, nous a déclaré, avec un brillant sens de la formule : « En biologie, ce qui était de la science-fiction il y a sept ans est aujourd'hui de la science. » J'ai été marqué par cette formule, par laquelle je tiens à conclure mon propos, car elle doit nous permettre de bien comprendre l'ampleur des enjeux qui s'ouvrent à nous depuis quelques années et qui animeront de nombreux débats à venir dans cet hémicycle. en séance, nous avons bien noté votre accord sur le fond, vos réserves sur la forme et surtout les avis de sagesse que vous avez donnés mercredi dernier sur les amendements de notre rapporteur ainsi que sur l'ensemble du texte.

L'enjeu est simple, et il est établi par l'Agence de la biomédecine depuis plusieurs années : le cadre législatif en vigueur pour les analyses génétiques à but médical n'a été pensé que dans le cas où la personne analysée est l'unique bénéficiaire des résultats de cet examen et des démarches médicales qui peuvent en découler. Est ainsi exclu le cas où la pathologie n'est pas détectée du vivant de la personne. lors, des familles subissant un décès en leur sein sont privées d'informations d'ordre génétique qui permettraient non seulement d'apporter des éléments complémentaires quant à la cause du décès, mais aussi et surtout d'engager des démarches de surveillance et de prévention auprès de proches potentiellement porteurs du gène en question.

conduit à ce que l'alinéa de l'article 16-10 du code civil relatif aux affaires de filiation protège de l'exhumation toute personne n'ayant pas expressément consenti à des analyses génétiques de son vivant. La société tout entière avait ainsi pris acte du fait que, dans les affaires de filiation, « la génétique devait s'arrêter à la porte des cimetières », selon l'expression alors employée par Jean-François Mattei. force est de constater que, si la proposition de loi soumise aujourd'hui à notre vote a bien trait à la génétique et au respect de la personne défunte, en aucun cas elle ne remet en cause les grands principes posés par nos lois de bioéthique. Tout d'abord, l'autorisation d'analyses génétiques n'est possible qu'à des fins de santé publique protégé le cadre que j'évoquais précédemment en matière de filiation. À cet égard, le présent texte ajoute dans la loi le cas où l'intérêt direct des analyses pour la santé n'est plus seulement celui de la personne analysée, puisqu'en l'occurrence elle est décédée, mais bien l'intérêt de ses ascendants, descendants et collatéraux.

ou dans le cadre d'une autopsie réalisée immédiatement après celui-ci. Votre décision présente le double avantage de couvrir la grande majorité, et même la quasi-totalité des situations, tout en évitant des dérives potentielles. L'intégrité du corps du défunt est bien respectée. concerne les personnes de la famille qui peuvent demander que l'on procède à ces analyses, je tiens à rappeler un point de vigilance quant aux termes, utilisés dans la proposition de loi, de « membres de la famille potentiellement cette rédaction ne respecte pas nécessairement les critères de rigueur scientifique et de précision juridique. Il m'aurait semblé plus prudent de préciser qu'il s'agit des membres potentiellement concernés sur le plan génétique, c'est-à-dire envers

potentiellement concernées sur le plan médical. Vous avez pris grand soin, d'une part, de préciser davantage encore les modalités de transmission de ces informations, qui peuvent être extrêmement lourdes de conséquences, notamment sur le plan psychologique, et, d'autre part, de consacrer le respect au droit à la non-information dont disposent les apparentés du défunt : on peut vouloir ne pas savoir si l'on est porteur d'anomalies génétiques ayant des conséquences sur la santé. santé. Mes chers collègues, ce texte répond à une forte demande de la part des professionnels concernés et des familles, et il s'inscrit dans la continuité des progrès techniques accomplis dans le domaine de la génétique à but médical.

Il comble une lacune sans toucher en rien l'édifice forgé par nos lois de bioéthique.

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, ce texte traduit, parmi bien d'autres, l'évolution de notre société contemporaine, en matière de science comme de moeurs. En effet, la génétique nous permet aujourd'hui d'analyser les caractères héréditaires familiaux prédisposant à la survenue de pathologies pour les descendants. Il s'agit de prévenir pour lutter contre les maladies aux caractères génétiquement transmissibles ; je pense non seulement au cancer, qui mine notre société, mais aussi à d'autres maladies, notamment dans le cadre du développement de la neurogénétique, de la cardiogénétique et de bien d'autres disciplines. L'état actuel de la technologie et les progrès de la science nécessitent une évolution législative, afin de mettre en adéquation ces progrès humains avec la réglementation en vigueur. C'est là une attention parfaitement légitime. La loi subordonne actuellement au consentement du patient les analyses génétiques, même lorsque celles-ci sont demandées par les descendants. Faute de ce consentement, ces analyses sont impossibles. Il convient donc de faire évoluer la loi et de la rendre compatible avec la pratique de ce qu'il est convenu d'appeler une médecine de précision. Le but est, naturellement,

Dans certains cas, ces analyses sont nécessaires, voire indispensables, pour établir les diagnostics les plus pertinents et, par là même, prescrire les traitements les plus appropriés. Grâce à ce dépistage précoce de la maladie, les oncogénéticiens pourront mieux informer les membres de la famille du défunt quant aux risques encourus et préconiser la meilleure surveillance médicale. Je suis donc persuadé de son bien-fondé, et je le suis d'autant plus que ce texte ne porte pas atteinte, selon moi, à la dignité de la personne humaine ou au respect de la vie privée.

me paraît plus positif que fâcheux. En effet, dans le rapport de synthèse remis hier, après plusieurs mois de travaux, figurent, parmi les neuf thématiques abordées, divers points qui soulèvent des polémiques- Michel Amiel en a parlé -pour des raisons plus philosophiques, religieuses ou politiques que purement scientifiques. Ces points de tension susciteront des débats qui auraient obéré l'avancée significative que permet notre proposition de loi. Or la sérénité permet d'être plus efficient. J'ose simplement espérer que ce texte fera rapidement partie de notre droit positif : ce serait là une avancée majeure, accomplie sans bruit ni effusion. Aujourd'hui, grâce à la recherche médicale, nous savons que 5 % des cancers surviennent chez des personnes présentant une prédisposition héréditaire. Ces tumeurs se développent souvent à des âges plus précoces, cinquante ans, et concernent plusieurs membres d'une famille. Si, dans une même famille, plusieurs personnes de la même branche, paternelle ou maternelle, ont été affectées par un cancer, une consultation oncogénétique oncogénétique est conseillée. Le but d'une telle consultation est donc d'évaluer s'il existe, dans une famille, un risque particulier de tumeur, ou si ce dernier peut être évité et expliqué par une prédisposition héréditaire. lors, il s'agit d'identifier les altérations génétiques héritées, qui peuvent induire un risque plus élevé de développer un cancer. Les progrès de la génétique permettent d'analyser les transmissions des caractères héréditaires prédisposant à la survenue de pathologies, notamment de cancers. À ce titre, il est parfois nécessaire de remonter le cours de l'histoire familiale, afin de conseiller les apparentés vivants il est nécessaire de recourir à des analyses sur des personnes décédées, afin d'obtenir des informations pouvant être utiles à la famille. Depuis plusieurs années, des analyses sont faites par prises de sang chez des patients ayant un risque élevé d'être porteurs d'une anomalie prédisposante. Ces prélèvements sont conservés longtemps, même si le patient est décédé. Il apparaît ainsi que les évolutions technologiques et les progrès scientifiques nécessitent une évolution législative : il convient de mettre en adéquation ces progrès et la réglementation. Les avancées concernent différents secteurs de la génétique, à l'instar de la cardiogénétique ou de la neurogénétique. On peut ainsi envisager tout un champ des possibles,

La loi actuelle impose le consentement du patient. Or, en l'espèce, ce consentement est par définition impossible à obtenir. Chacun l'a compris, cette proposition de loi ne tend évidemment pas à porter atteinte à la dignité de la personne ni à attenter au respect de la vie privée.

À l'instar des maillons ADN qui constituent la chaîne génétique de l'individu, l'individu constitue un maillon de la chaîne familiale. Tout l'enjeu réside donc dans la nécessité de concilier liberté de l'individu et inscription dans l'histoire de l'héritage génétique familial. En renforçant le traitement précoce des différentes strates de l'arbre généalogique, cette proposition de loi permet de renforcer sa vitalité. un écrivain de ma région, Frédéric Mistral, « les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut », les progrès de la science, conjugués aux dispositions de ce texte, permettent d'ajouter à la hauteur de l'arbre l'épaisseur des branchages, qui, grâce au traitement précoce, pourront poursuivre leur développement ! Je vous remercie

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian, du 2 juillet 1962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

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est des mesures qui font consensus, mais qu'aucun gouvernement, une fois arrivé au pouvoir, ne met en oeuvre. L'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie après l'indépendance de ce pays en fait partie. Je salue donc l'initiative de notre collègue Dominique de Legge, à laquelle nous sommes nombreux, sur toutes les travées de cet hémicycle, à nous être associés. Cette proposition de loi répond à une demande récurrente du monde combattant, mais systématiquement rejetée par les gouvernements successifs. Elle met un terme à une situation d'injustice criante, souvent dénoncée au Sénat. La carte du combattant manifeste la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l'ont servie par les armes. Elle ouvre droit à des avantages symboliques, comme le port de la croix du combattant, ou matériels, notamment le bénéfice d'une retraite annuelle d'environ 750 euros et d'une demi-part fiscale supplémentaire. Créée à la suite de la Première Guerre mondiale, cette carte a été étendue aux conflits ultérieurs, parfois même avant qu'ils ne soient terminés. En 1993, elle a été attribuée aux soldats de la quatrième génération du feu, qui ne participent plus à des guerres à proprement parler, mais à des opérations extérieures. Néanmoins, la reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires, bien souvent de jeunes appelés, qui ont participé à ce qui était désigné comme des « opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord », a été plus difficile. Un titre de reconnaissance nationale qui n'ouvre droit ni à la retraite du combattant ni à la demi-part fiscale a tout d'abord été créé en 1967. En 1974, la carte du combattant a finalement été attribuée, mais uniquement aux militaires ayant servi jusqu'au 2 juillet 1962, date de l'accès à l'indépendance de l'Algérie. Cette date est certes postérieure au cessez-le-feu du 18 mars, mais elle ne correspond pas pour autant à la fin de la présence militaire française sur ce territoire. En effet, en application des accords d'Évian, le retrait s'est fait de manière progressive jusqu'au 1 juillet 1964. Au total, plus de 75 000 soldats français ont été déployés pendant cette période. En 1999, le législateur a reconnu que les événements d'Afrique du Nord étaient une guerre, et que cette dernière avait pris fin avec l'accès de l'Algérie à l'indépendance. Les militaires français présents sur le sol algérien après cette date ne participaient donc pas à une guerre. Toutefois, leur présence est tout à fait assimilable à une opération extérieure. Dès lors, on voit mal ce qui s'oppose à la reconnaissance de leur qualité de combattant. Je précise que certaines des OPEX reconnues par l'arrêté du 12 janvier 1994, texte modifié plusieurs fois, étaient moins intenses et moins dangereuses que la présence en Algérie entre 1962 et 1964. Il s'agit donc d'une question d'équité entre générations du feu. Il s'agit également d'une question d'égalité entre frères d'armes. En créant ce que l'on appelle communément la « carte à cheval », la loi de finances pour 2014 a en effet instauré une différence de traitement assez injustifiable. Un soldat présentant quatre mois de service, arrivé en Algérie le 30 juin 1962, a ainsi droit à la carte du combattant et aux avantages y afférents, alors que son compagnon d'armes arrivé le 3 juillet en est privé. La question budgétaire ne saurait être un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. Le nombre de bénéficiaires potentiels est inférieur au nombre de titulaires de la carte du combattant qui décèdent chaque année. Le coût sera appelé à se réduire rapidement au cours des prochaines années, compte tenu de la démographie des anciens combattants. Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, Mme la secrétaire d'État aux anciens combattants s'est engagée à mener un travail sur la question, et notamment à évaluer le coût Il semble que ce travail ait abouti, puisque le Premier ministre a annoncé, quelques jours avant l'examen en commission du présent texte, l'intention du Gouvernement de mettre en oeuvre cette mesure. En commission, Mme Geneviève Darrieussecq nous a suggéré d'attendre le prochain projet de loi de finances. J'entends cette demande et je serais le premier à me réjouir si le Gouvernement venait à mettre en oeuvre cette mesure par voie réglementaire avant l'aboutissement de cette proposition de loi. dans l'immédiat, je vous propose néanmoins de réaffirmer clairement la volonté du Sénat d'accorder aux anciens combattants la reconnaissance que nous leur devons et d'adopter ce texte, qui a recueilli l'unanimité en commission, signe du consensus qui existe parmi nous ! La parole

tout particulièrement aujourd'hui. Ce débat montre l'intérêt que toute la représentation nationale et la classe politique en général portent à ceux qui ont eu l'honneur de servir la France. Nous sommes réunis pour étudier une proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie sur la base des accords d'Évian. Comme vous le savez, c'est là une disposition que le Gouvernement soutient sur le fond : ma collègue Geneviève Darrieussecq vous a indiqué que cette mesure serait présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français de cette époque furent en effet déployés sur ce territoire entre les mois de juillet 1962 et de juillet 1964, à la suite des accords d'Évian. Malheureusement- nous dressons avec vous ce constat -, ils n'ont jamais pu bénéficier de la carte du combattant et des avantages qui s'y attachent.

Toutefois, ils n'ont pas droit à la carte du combattant. Dans le cadre de la loi de finances du 29 décembre 2013, pour 2014, les conditions d'attribution de la carte du combattant ont été étendues aux personnes présentes en Afrique du Nord au-delà de la date du 2 juillet 1962, à condition que leur séjour ait commencé avant cette date

Cette décision fait suite à un travail d'échanges et de concertation intense. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, par la voix de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq, le Gouvernement s'est engagé à étudier l'ensemble des demandes du monde combattant. Dans ce cadre, lors de ses déplacements dans toute la France, Mme Darrieussecq a eu l'occasion de rencontrer près de trente délégations départementales pour discuter de leurs attentes. Par ailleurs, sous sa présidence, le ministère des armées a constitué trois groupes de travail, qui ont mené près de vingt réunions avec les représentants des associations d'anciens combattants et ont permis d'étudier vingt-huit sujets différents.

Ce travail inédit a permis d'évaluer précisément l'opportunité, la faisabilité juridique et technique ainsi que les coûts de ces différentes demandes.

Dans le respect de cette méthode et de ce calendrier, Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont proposé au Premier ministre d'inscrire cette mesure dans le prochain projet de loi de finances. Pour aboutir à cette décision, le ministère des armées a mené une étude approfondie des effectifs présents en Algérie à cette époque. Un travail statistique poussé, sur la base des données dont dispose le service historique de la défense, le SHD, a donc été consacré aux dispositifs français présents en Algérie à cette époque : les plans « Chartres » successifs, la concession de la base de Mers el-Kébir et celle des bases d'essais situées au Sahara. étude, à ne pas prendre en compte le public déjà éligible à la carte du combattant dans le cadre du dispositif dit « à cheval » ; à ne pas comptabiliser deux fois les effectifs d'un dispositif affecté pour un emploi dans un autre dispositif ; et à se concentrer sur les effectifs d'appelés, qui, à la différence des engagés, ne sont pas susceptibles de déjà détenir la carte du combattant au titre d'un autre conflit. Ces travaux ont permis d'aboutir à l'estimation d'un effectif cumulé de 75 319 appelés ayant été déployés en Algérie entre le mois de juillet 1962 et celui de juillet 1964. À partir des données statistiques d'évolution démographique, il y aurait, en 2019, un total de 49 819 bénéficiaires potentiels d'une carte du combattant d'Algérie 1962-1964. Compte tenu de leur âge, ces bénéficiaires sont en droit de percevoir la retraite du combattant. Les modalités de versement de cette prestation conduisent à évaluer le coût budgétaire prévisionnel à 37 millions d'euros environ, si l'on prend en compte tous les demandeurs potentiels, ou à 30 millions d'euros en moyenne en année pleine. S'y ajoute de façon indirecte le coût fiscal associé, qui est, lui aussi, estimé à 30 millions d'euros annuels par les services du ministère de l'action et des comptes publics. L'extension envisagée pour la période 1962-1964 sera menée à législation constante, sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, cet article permet l'attribution de la carte du combattant au titre de « la participation à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ». de l'attribution de la carte est possible, puisque les accords d'Évian du 18 mars 1962, en vertu desquels les militaires français ont servi en Algérie après 1962, peuvent être regardés comme relevant des engagements internationaux de la France. L'article L. 311-2 renvoie à un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget pour la détermination des périodes à prendre en compte pour chacune des opérations ou chacune des missions concernées. Ainsi, cette extension sera rendue possible en modifiant ledit arrêté, qui date du 12 janvier 1994, sans qu'il soit opportun de passer par une loi qui, au total, pourrait compliquer l'application de la mesure. de la mesure. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, au regard des éléments que je viens de vous exposer brièvement, vous admettrez que cette proposition de loi ne présente plus de nécessité en l'état

Toutefois- j'insiste sur ce point -, votre proposition de loi va dans le sens de l'action du Gouvernement, et nous nous en félicitons. Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour l'examen du projet de budget par la Haute Assemblée : nous ne doutons pas une seule seconde de votre plein et entier soutien à cette disposition du futur budget. Ah ! Je vous remercie vivement de votre attention et de votre intérêt, qui est aussi celui du Gouvernement, pour le monde combattant. La parole

au cours du siècle dernier, la France a dû panser les plaies des grands conflits qui l'ont successivement minée. Aujourd'hui encore, à côté du devoir de mémoire, nous poursuivons le travail de réparation à l'égard de toutes celles et de tous ceux que l'histoire a emportés dans ses tourments. La carte du combattant, par les droits qui lui sont attachés, constitue le principal vecteur de la reconnaissance de la Nation envers les anciens combattants. les anciens combattants. Pensée en 1926 pour la première génération du feu de la Grande Guerre, elle a été progressivement étendue jusqu'à concerner une deuxième, puis une troisième et enfin une quatrième génération du feu de soldats engagés les opérations extérieures. Nous sommes tous très attachés à la mise en oeuvre constante par l'État de la reconnaissance des sacrifices endurés par les militaires de carrière, par les appelés et par les supplétifs. Pour autant, nous n'ignorons rien des quelques imperfections de ce régime de reconnaissance, en particulier de l'iniquité qui perdure parfois au sein de certains de ses dispositifs. Il revient au législateur de les corriger. Comme vous le savez, mes chers collègues, la spécificité des conflits issus des indépendances a rendu plus tardive la reconnaissance du droit à réparation pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Il aura en effet fallu attendre 1974, soit douze ans après les accords d'Évian, pour que les militaires et les appelés accèdent clairement au statut d'ancien combattant et bénéficient enfin de la carte du combattant. Comment pouvait-il en être autrement ? Malgré les combats, malgré les souffrances, malgré les sacrifices, il n'a été question pendant longtemps que « d'opérations effectuées en Afrique du Nord a été effacé par la loi du 18 octobre 1999, qui a reconnu la qualification de guerre d'Algérie. Nous le devions

d'Évian. Malheureusement, 535 soldats français ont été tués sur un territoire, où, malgré le cessez-le-feu, les horreurs ont continué. Je pense notamment au terrible massacre d'Oran, le 5 juillet, et je refuse d'oublier le sort tragique des harkis. Face à tout cela, le groupe du RDSE considère comme un devoir l'attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964. L'adoption de la proposition de loi rétablirait une égalité de traitement entre les différentes générations du feu, mais aussi entre les frères d'armes, car la carte dite « à cheval », bien que légitime et attendue, avait introduit une nouvelle injustice. De plus,

Mes chers collègues, pendant longtemps, les parlementaires ont connu des débats passionnés, s'agissant de la guerre d'Algérie. Il faut dire que ce conflit n'opposait pas seulement deux peuples- les Français aux Algériens -, mais aussi les Algériens aux Algériens et les Français aux Français. Certains d'entre nous ont vécu au plus près cette période tragique. Aujourd'hui, le temps et le travail de mémoire ont fait oeuvre d'apaisement. C'est donc dans la sérénité que nous pouvons approuver

notre nation va enfin accorder à ces combattants la reconnaissance symbolique et financière à laquelle ils aspirent bien légitimement. Comme l'a rappelé dans son rapport notre collègue Philippe Mouiller, dont je salue de nouveau le travail, cette revendication s'est heurtée durant de trop nombreuses années à des obstacles politiques et budgétaires, de sorte que nous réparons aujourd'hui une longue injustice, grâce à cette proposition de loi

Sans cette volonté présidentielle et gouvernementale, mes chers collègues, le texte que nous votons aujourd'hui n'aurait probablement pas porté ses fruits, à l'image de ses prédécesseurs. Cela doit être souligné Notre groupe, qui a soutenu sans faille cette revendication auprès de Mme la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, se félicite de la voir aboutir et votera ce texte, qui sera pleinement satisfait par la prochaine loi de finances. À l'occasion de ce vote,

attentive, afin d'identifier précisément les priorités et les urgences. En l'occurrence, cette méthode de travail a permis d'affiner le chiffrage, par les services de l'État, de la mesure d'équité que nous adoptons aujourd'hui, puis d'en sécuriser le financement auprès du Premier ministre. Il était de sa responsabilité de procéder ainsi, tout comme le Parlement est entièrement dans son rôle en déposant et en discutant une proposition de loi Il est heureux que les deux démarches aient enfin convergé au bénéfice des anciens combattants. Rendez-vous est donc pris pour le prochain débat budgétaire ! La parole

Cette date concerne les engagés en Algérie comme en Tunisie et au Maroc. Pourtant, si la fin de la guerre d'Algérie est officiellement fixée à la signature des accords d'Évian et l'indépendance algérienne au 2 juillet 1962, le contingent français est resté sur zone jusqu'en 1964. étaient présents au 2 juillet 1962, 103 000 en janvier 1963 et encore 50 000 en juillet 1964. En outre, 535 soldats français sont morts en Algérie après l'indépendance et le début du retrait des troupes.

anciens combattants, présents en Algérie à cheval sur les deux périodes- avant et après le 2 juillet 1962 -, de faire valoir leur droit à reconnaissance. Les dispositions prévues dans cette proposition

toujours pas accordé aux militaires français déployés en Algérie entre 1962 et 1964 ? Ceux qui ont perdu la vie pendant cette période ont droit à la qualification

Nous sommes face à une aberration : celui qui est arrivé sur place le 1 juillet 1962 a pu obtenir la carte du combattant, alors que celui qui est arrivé le 3 juillet 1962 n'a pu en bénéficier. Pourtant, vous en conviendrez, ces deux personnes se trouvaient dans le même peloton et y ont effectué, ensemble, les mêmes missions, les mêmes jours, aux mêmes horaires. Je souhaite préciser qu'il ne s'agit ici en aucun cas de réécrire

en Algérie. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, plusieurs amendements avaient été déposés en ce sens. À l'époque nous nous étions heurtés à un refus du Gouvernement, qui nous demandait du temps.

Je suis ravie de soutenir cette avancée concrète, à laquelle je me suis jointe en cosignant ce texte. Baignant dans un environnement familial militaire, je ne saurais rester insensible à cette demande si légitime. légitime. Je poursuivrai mes propos en évoquant le dénominateur commun qui nous unit aujourd'hui : la République. Nous tous ici croyons en la République de l'égalité et de la justice, en la République de la dignité. ici, nous défendons l'expression de la reconnaissance de la Nation envers ses combattants d'hier et d'aujourd'hui, tous, sans la moindre distinction ! Ainsi, ne pas permettre aux soldats ayant combattu en Algérie après 1962 de bénéficier de la carte du combattant, contrairement aux militaires français engagés au Maroc ou en Tunisie après les indépendances de ces pays, est une inégalité. Les oublier est une injustice, ignorer leur sacrifice et leur courage, une profonde indignité. De plus, il ne s'agit pas de travestir l'histoire, mais de rétablir des faits. Si les accords d'Évian entendent instaurer le cessez-le-feu et la fin de la guerre d'Algérie, alors les opérations de sécurité conduites entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964 l'ont été dans le cadre d'opérations extérieures. Est-il vraiment utile de rappeler, mes chers collègues, que le titre de reconnaissance de la Nation, qui, par nature, marque la participation à un conflit armé comportant un risque d'ordre militaire, est attribué aux soldats En outre, je veux croire, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement demeure sensible à cette cause. En effet, je me souviens de l'intervention de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des armées, à l'occasion de la discussion de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » au mois de décembre dernier, ainsi que de son sens de l'écoute. Je la crois imprégnée de sincérité et de la ferme volonté de faire avancer ce douloureux dossier. L'annonce de l'inscription de cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2019 confirme ses propos, et nous saluons cet engagement. C'est la première fois qu'un gouvernement va jusqu'au bout en donnant satisfaction à cette demande ; il est important de le souligner. Cependant, il y a urgence. Le temps est compté. N'attendons pas la disparition des derniers soldats pour enfin prendre en considération ce qu'ils demandent depuis tant d'années. d'années. Ils ont tout donné, parfois même jusqu'au dernier souffle, ils méritent notre reconnaissance, ils méritent le bénéfice de la carte du combattant. Reconnaître l'action de nos anciens, c'est aussi l'honneur de notre pays. Ils sont la France.

D'une certaine manière, ce texte participe à cet exercice. Mes chers collègues, n'oublions pas ces noms, ces visages, ces vies consacrées. C'est pourquoi le groupe Union Centriste apporte tout son soutien à cette proposition de loi déposée par Philippe Mouiller et la votera. La parole est à

pour explication de vote. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour trouver une issue favorable à une demande qui a souvent occupé nos débats ces dernières années, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, autour de propositions de loi émanant de tous les bancs. C'est ce travail parlementaire que je veux d'abord saluer, qui va finalement aboutir et permettre de répondre à une sollicitation récurrente des associations d'anciens combattants, telles que l'UNC, la FNACA et d'autres, dont j'ai l'habitude de côtoyer les représentants dans mon département, le Calvados. Oui, nous allons réparer une inégalité persistante entre soldats français, selon qu'ils ont été engagés en Algérie avant ou après le 2 juillet 1962 ! Dans les faits, l'indépendance de l'Algérie n'a nullement signifié le départ immédiat de nos troupes du territoire algérien. 1962 et 1964, plusieurs dizaines de milliers de soldats français y étaient toujours présents et 535 d'entre eux y ont trouvé la mort. La présente proposition de loi permet de considérer cette période non pas comme un temps de guerre, mais comme un moment pouvant relever de la caractérisation d'opérations extérieures, au bénéfice de la carte du combattant. Rappelons que cette dernière, qui manifeste la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l'ont servie par les armes, permet de bénéficier d'avantages symboliques, comme le port de la croix du combattant, ou d'avantages matériels : une retraite annuelle de près de 750 euros et une demi-part fiscale supplémentaire. Les soldats qui ont été engagés en Algérie avant comme après le 2 juillet 1962 y ont bien évidemment droit. Il y va de l'équité entre frères d'armes et, au-delà, de l'égalité entre générations du feu. Chaque quinquennat connaît des avancées en faveur du monde combattant. Je me félicite donc de la décision récemment annoncée par le Gouvernement d'octroyer, à partir de 2019, la carte du combattant aux soldats français déployés en Algérie après le 2 juillet 1962. Selon le Gouvernement, cela concernerait potentiellement 50 000 bénéficiaires. Je m'étais moi-même fait la porte-parole de leur légitime demande de reconnaissance lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 et, encore plus récemment, le mois dernier, lors de l'audition de Mme Darrieussecq par le par le groupe d'études Sénateurs anciens combattants et de la mémoire combattante, dont je suis membre. Je voudrais terminer mon propos en rappelant que beaucoup de choses ont été faites en direction du monde combattant lors du dernier quinquennat,

la refonte des aides sociales de l'ONACVG ou encore le travail mémoriel souhaité par le Président François Hollande, lequel a multiplié les signes forts. Toutes ces actions méritent d'être saluées. Le groupe socialiste votera ce texte, comme une nouvelle main tendue à ces anciens soldats et pour les assurer que la France ne les oublie pas. Nous voterons cette proposition de loi également pour saluer le rôle du Parlement et souligner son travail, particulièrement sur ce sujet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues de Legge et Mouiller fait oeuvre de justice et de bon sens. Elle répond à une demande des associations d'anciens combattants et répare une inégalité persistante entre militaires français, selon qu'ils ont été engagés en Algérie avant ou après le 2 juillet 1962. Comme cela a été rappelé, 50 000 d'entre eux étaient encore présents sur le territoire algérien en 1964 et 535 ont perdu la vie après l'accès de l'Algérie à l'indépendance.

Les désaccords entre certaines associations ont été levés, et le monde combattant est maintenant unanime. Pourtant, les gouvernements successifs ont refusé d'accéder à leurs demandes. Pourquoi ?

Cette mesure coûterait 37,5 millions d'euros au titre de la retraite du combattant et entraînerait une dépense fiscale que l'on peut évaluer à 30 millions d'euros au titre de la demi-part fiscale, soit une dépense totale de 70 millions d'euros. Reconnaissons que, face aux dépenses abyssales, passées ou à venir,

Le Président de la République a eu des mots justes lors de sa visite en Algérie en décembre dernier : il ne faut rien renier du passé, n'avoir aucun tabou, mais regarder vers l'avenir d'une relation assainie assainie et refondée. Cette proposition de loi permet de reconnaître symboliquement une dimension de notre passé commun, qui doit enfin être assumée pour être dépassée. Les oppositions sont donc aujourd'hui levées. Nous sommes entrés dans l'ère du consensus. Nous sommes heureux de constater que ce consensus est désormais partagé par le Gouvernement.

Le Gouvernement souhaite désormais inscrire cette disposition dans le prochain projet de loi de finances. Ce choix courageux était attendu depuis plusieurs années. Notre groupe salue donc le respect de la parole donnée et la volonté d'avancer avec toutes les parties prenantes : parlementaires, associations et anciens combattants. Cette proposition de loi n'en est que plus importante. Elle constitue une étape bienvenue sur la route de la reconnaissance de nos anciens combattants,

alors que nous nous apprêtions à débattre en commission de notre texte, le Gouvernement annonçait le financement de cette mesure dans le prochain budget et concluait qu'il n'y avait plus lieu de débattre,

La méthode, un peu grossière, n'est pas nouvelle : elle a été utilisée pour de nombreux textes d'initiative sénatoriale, qui furent ainsi purement et simplement récusés à l'Assemblée nationale pour renaître sous une forme sensiblement identique, mais, cette fois, sur l'initiative du Gouvernement. Je souhaite rappeler ici que, depuis 2008, la Constitution prévoit un ordre du jour partagé, accordant une place à l'initiative parlementaire. Je ne peux que déplorer

l'intérêt. Elle n'augure pas bien de l'état d'esprit du Gouvernement dans la perspective de la réforme constitutionnelle, dont on perçoit qu'elle ne va pas dans le sens d'un renforcement des droits et du pouvoir du Parlement.

sa mémoire et la reconnaissance due à ceux qui ont risqué ou perdu leur vie pour elle, se réduise pour le Gouvernement à une simple question comptable. Je remercie le rapporteur Philippe Mouiller et le président de la commission Alain Milon d'avoir maintenu ce texte. Il nous a paru important de rendre justice à ces combattants et d'honorer par là même la mémoire de leurs frères tombés en Algérie durant cette période. Je dis « nous car cette proposition de loi a recueilli plus de 120 signatures issues de toutes les formations politiques, pour exprimer de manière solennelle, par la voix des représentants de la Nation, notre reconnaissance à ces combattants injustement écartés d'une prestation à laquelle ils avaient droit.

La séance est reprise. affaires européennes, de la proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 du règlement, en faveur de la préservation d'une Politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires, présentée par M. Daniel Gremillet, Mme Pascale Gruny, MM. Claude Haut et Franck Montaugé

Dès juillet 2017, avec Daniel Gremillet, Claude Haut et Franck Montaugé, nous avons ainsi publié un rapport d'information intitulé,

Au regard des éléments préparatoires publiés par les instances européennes et des positions prises par les autorités françaises, il nous a semblé indispensable de revenir sur le sujet. En effet, l'architecture de la réforme en gestation est manifestement éloignée de nos recommandations. Compte tenu de l'importance capitale de la PAC, le Sénat ne pouvait naturellement pas en rester là. La seconde proposition de résolution européenne, qui a été adoptée à l'unanimité le 19 avril dernier par notre commission des affaires économiques et notre commission des affaires européennes, confirme et prolonge nos réflexions antérieures. Nous voulons une PAC forte, rénovée et répondant aux attentes des agriculteurs. Je ne peux manquer de m'émouvoir de l'ampleur de la baisse annoncée pour les moyens budgétaires de la PAC. La Commission européenne « communique » sur une diminution de 5 % en euros constants. En prenant en compte l'inflation, la diminution réelle atteindrait 15 %. S'y ajouterait aussi l'impact, mécaniquement défavorable à la France, de la poursuite du processus de convergence des paiements directs à l'intérieur de l'Union européenne au bénéfice des nouveaux membres. Je me suis aussi inquiétée à la lecture des propositions pour la future PAC 2021-2027 publiées le 1juin par la Commission européenne. Ces dernières reposent reposent sur quatre grandes orientations. La première concerne le nouveau mode de mise en oeuvre imaginé pour la PAC. Concrètement, l'approche uniforme serait remplacée par davantage de subsidiarité : des plans stratégiques seraient élaborés par les États membres, puis validés par la Commission. Commission. Ce est supposé simplifier le coeur de la politique agricole commune en retenant une approche par les résultats plutôt que par les moyens. Il présente néanmoins un double risque de « renationalisation » et de distorsion de concurrence. La deuxième orientation de la nouvelle PAC vise à établir des conditions plus équitables grâce à un meilleur ciblage des aides. En résumé, les paiements directs aux agriculteurs seraient réduits jusqu'à 60 000 euros et plafonnés à 100 000 euros par exploitation en déduisant les coûts de main-d'oeuvre. La troisième orientation tend à encourager l'innovation et la recherche. Ainsi, 10 milliards d'euros issus du programme Horizon y seraient affectés. La dernière orientation défendue par la Commission a pour objet de relever les ambitions environnementales et climatiques de la PAC. Les paiements directs seraient ainsi subordonnés à des exigences accrues : au-delà du « verdissement » actuel considéré comme acquis, il y aurait à l'avenir treize exigences réglementaires- à commencer par les directives Nitrates, Bien-être animal, Habitat, Oiseaux -auxquelles s'ajouteraient douze conditions agroenvironnementales définies au niveau européen, dont cinq nouvelles. Les États membres ou les régions auraient ensuite à préciser aux agriculteurs les règles à suivre pour mettre en oeuvre ces grands principes.

En définitive, la dernière des quatre orientations annoncées le 1 juin représente à l'évidence une innovation importante dont il faudra prendre le temps de mesurer l'impact. En première analyse, la question posée est celle de la nature même de la PAC : s'agira-t-il toujours à l'avenir d'un budget de soutien à une activité économique ou bien cette politique deviendra-t-elle un budget d'accompagnement de la réglementation environnementale ? La parole

j'axerai mon propos sur la comparaison entre l'économie générale de notre proposition de résolution européenne et le contenu des propositions législatives de la Commission européenne, dont ma collègue Pascale Gruny vient de vous présenter la synthèse. D'une façon générale, les réflexions de la Commission européenne, censées préfigurer les contours de la prochaine réforme, sont assurément décevantes à plusieurs titres. En effet, elles ne reprennent que très imparfaitement, voire contredisent sur le plan budgétaire, aussi bien les recommandations de la première résolution du Sénat du 8 septembre 2017 que celles de notre nouvelle- et seconde -proposition de résolution européenne sur la PAC. J'observe toutefois que les négociations ne font que commencer. Par ailleurs, les autorités françaises ont d'ores et déjà jugé « inacceptables » les propositions de la Commission européenne au titre des crédits budgétaires de la PAC pour la période 2021-2027 dans le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Nous attendons donc désormais avec intérêt, monsieur le ministre, de connaître la position du Gouvernement sur le contenu même des propositions formulées par la Commission européenne. Dans cette perspective, le seul énoncé des quatre orientations avancées par la Commission européenne, à savoir la confirmation du nouveau mode de mise en oeuvre de la PAC, le ciblage des aides, l'encouragement de la recherche et l'approfondissement des ambitions environnementales, apparaît sensiblement différent de nos propres priorités. Pour mémoire, la proposition de résolution européenne du Sénat met en avant les cinq points suivants : premièrement, l'impérieuse nécessité d'un budget stable en euros deuxièmement, de vives inquiétudes et réticences à l'égard du nouveau mode de mise en oeuvre envisagé de la PAC ; troisièmement, le refus du en matière de règles de concurrence et de gestion de crise quatrièmement, la réaffirmation des préconisations antérieures en matière de commerce international ; enfin, de fortes interrogations sur la possibilité d'aboutir à un accord sur la PAC d'ici au printemps 2019. Au total, le texte de notre nouvelle proposition de résolution européenne comporte vingt-trois demandes et recommandations, précédées par un ensemble de quatre considérants. Il a vocation à compléter notre première proposition de résolution européenne, adoptée par le Sénat le 8 septembre 2017. Il reprend d'ailleurs explicitement et sans aucun changement la partie de cette résolution relative au commerce international, cette reprise étant justifiée par l'importance des négociations commerciales en cours, à commencer par celles avec les pays du MERCOSUR, qui ont dominé l'actualité des derniers mois. Mes collègues rapporteurs insisteront dans quelques instants sur certains points clés des propositions législatives de la Commission européenne avec laquelle nous avons des divergences plus ou moins importantes. Permettez-moi cependant de conclure mon propos sur une note positive- il en faut une ! La Commission européenne prévoit en effet d'allouer un minimum de 2 % de la dotation en paiement direct au soutien de l'installation des jeunes agriculteurs. Sur ce point capital, comme d'ailleurs sur la recherche et l'innovation, nos préoccupations ont été prises en compte. En définitive, monsieur le ministre, nous avons grandement besoin que la France continue à exprimer une volonté politique forte pour soutenir la politique agricole commune, car, pour reprendre les termes du commissaire Phil Hogan, « jamais cette politique n'a été autant sous pression ».

la politique agricole européenne est à un tournant historique, peut-être plus important encore que celui qu'elle a connu dans les années 1990. Véritable politique fondatrice de l'Union européenne, elle en est depuis les années soixante le volet le plus intégré. Or c'est justement à l'heure où l'on parle d'une Europe en crise que la Commission européenne a délibérément choisi de sacrifier sa politique la plus européenne. Plus qu'une faute, c'est un véritable renoncement. En proposant de réduire le budget de la politique agricole commune de plus de 40 milliards d'euros pour la prochaine période du cadre financier pluriannuel allant de 2021 à 2027, la Commission européenne a suscité l'indignation du monde agricole. Ces chiffres, déjà très préoccupants, sont malheureusement présentés sous leur meilleur jour. Compte tenu de l'inflation que la Commission ignore volontairement, la baisse du budget de la politique agricole commune sera davantage de l'ordre de 12 % que des 5 % annoncés. Les subventions directes seront sévèrement touchées par une coupe brutale de 8 %. Le deuxième pilier de la politique agricole commune, qui permet des investissements dans des projets d'avenir ruraux serait quant amputé d'un quart de son budget par rapport à la période précédente. Pour la France, cela entraînera concrètement une réduction de plus de 600 millions d'euros par an des aides directes de la PAC. Cela se traduira instantanément par une coupe sèche dans les revenus des agriculteurs. Comment peut-on le permettre, alors qu'un tiers des agriculteurs français ont des revenus très faibles ? Il est d'ailleurs paradoxal pour un gouvernement français de défendre au niveau national une meilleure rémunération pour les agriculteurs dans un projet de loi que nous aurons à connaître d'ici à la fin du mois de juin, tout en laissant, au niveau européen, opérer des baisses drastiques et directes des revenus des agriculteurs. Le commissaire européen Phil Hogan, décrivant ces perspectives budgétaires, a parlé d'un « résultat très équitable pour les agriculteurs ». Permettez-moi de lui répondre que, au regard de la situation de notre agriculture, ces paroles sont inacceptables, incroyables de la part du commissaire de la part du commissaire qui doit porter le projet de l'agriculture et de l'agroalimentaire au sein de l'Union européenne. Il n'est pas question de contester la complexité de l'équation financière que la Commission européenne doit résoudre en établissant son cadre financier pluriannuel. Au regard de ses ambitions, l'Union européenne n'a pas assez de ressources. Or, tout en constatant que la perspective du Brexit ampute potentiellement son budget de 12 milliards d'euros, l'Union européenne aspire à accroître ses ambitions en répondant à de nouvelles priorités politiques, notamment en matière de défense ou de migrations. Il est en revanche de notre devoir de dénoncer le fait que la Commission européenne finance ses nouvelles priorités en sacrifiant la PAC. On aurait pu imaginer une ambition budgétaire européenne bien plus forte tout en partant du socle de base, qui était la politique agricole commune. Cela donne l'amère impression que la Commission européenne la considère comme une vieille politique destinée à être abandonnée peu à peu. Croire cela, c'est témoigner d'une absence totale de vision à long terme. La politique agricole commune est, mes chers collègues, la condition première de la souveraineté de l'Union européenne. Elle permet d'assurer l'indépendance et la sécurité alimentaires de tout un continent. C'est pourquoi elle revêt des enjeux géostratégiques essentiels au XXIsiècle. Tous les autres grands pays l'ont compris. Les efforts budgétaires en matière agricole des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie ont considérablement augmenté ces dernières années, avec de véritables perspectives et de véritables ambitions. L'Union européenne s'apprête à faire l'inverse. C'est vrai ! Si une telle réduction du budget venait à être décidée, il s'agirait d'un revirement brutal, totalement à contre-courant de la politique suivie par les autres puissances mondiales. Face à cette situation, la France doit être ferme la France doit être ferme et intraitable, monsieur le ministre. Le Gouvernement doit être à la hauteur des enjeux. Les négociations préalables ont été un échec. Il n'est pas trop tard pour changer la donne. Mes chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Cela dépasse de loin nos appartenances politiques. Il s'agit de l'avenir de l'agriculture. Il s'agit de l'avenir de la ferme France. Il s'agit de l'avenir de nos territoires. Il s'agit d'assurer aux générations futures la garantie alimentaire. Le Sénat, au travers de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires européennes, s'est mobilisé depuis l'année dernière, pressentant des négociations délicates tant sur la nouvelle architecture de la politique agricole commune que sur son budget. Sur ce point, la proposition de résolution européenne appelle au strict minimum que la PAC bénéficie pour la période 2021-2027 d'un budget d'un montant stable en euros par rapport à la période précédente. Je vous invite donc à l'adopter, afin d'envoyer un signal fort à la fois au Gouvernement et aux institutions européennes. Très bien

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la réussite d'une réforme ne se mesure pas qu'à l'aune du budget qui lui est consacré, mais tout de même

Dans de telles conditions, ce que la loi qui fait suite aux états généraux de l'alimentation pourrait hypothétiquement faire gagner aux producteurs français, la PAC leur enlèverait, et peut-être même au-delà. Je ne le souhaite pas, bien entendu, mais je crois que nous avons un devoir de lucidité. Les propositions que nous faisons dans ce texte n'en sont donc que plus pertinentes. J'en reprendrai quelques-unes qui illustrent la responsabilité et la solidarité dont nous devons faire preuve à l'égard des acteurs du monde agricole, en premier lieu Le système du pur libre marché, qui place directement et en permanence le producteur seul face à des marchés volatils ou des acheteurs concentrés, est peu compatible avec une économie agricole variée, performante et durable. Les crises nombreuses doivent pouvoir faire l'objet d'interventions avec de nouveaux outils- je pense aux mécanismes contracycliques ou aux aides volontaires à la gestion des volumes du marché, comme le VCI, le volume Nous en appelons aussi à l'activation en temps opportun de la réserve européenne de crise et à sa gestion par période triennale. Les outils assurantiels et les fonds de mutualisation de gestion des risques doivent également être promus et accompagnés. Sur le plan des principes de gestion de la PAC, nous en appelons au pragmatisme pour être efficaces dans la concurrence et dans la gestion des crises nombreuses. À cet égard, la façon dont la France et l'Europe gèrent la révision de la carte des zones défavorisées simples est un contre-exemple absolu en matière de pragmatisme. Exactement ! Dans mon département,

1 million d'euros de perdus sur un total de 6 millions dans le Gers, terre ancestrale de polyculture et d'élevage. Stop au darwinisme agricole et au sacrifice délibéré des paysans les plus modestes Après des cas comme celui-là, injustifiables, inexplicables aux hommes et aux femmes qui en sont les victimes, il ne faut pas s'étonner que l'idée européenne régresse et que le populisme de rejet des grandes constructions de l'après-guerre gagne du terrain au péril de la démocratie.

proposition de résolution européenne. C'est pourquoi nous faisons des propositions qui vont dans le sens d'une meilleure insertion et d'une meilleure prise en compte des agriculteurs dans les diverses transitions auxquelles notre société et nos territoires doivent contribuer. Dans le cadre de la politique énergétique nationale et de la programmation pluriannuelle de l'énergie à venir, la PAC doit faciliter les investissements des agriculteurs en matière de production d'énergies renouvelables. Les cultures et les forêts stockent, on le sait, d'énormes quantités de carbone, et le pouvoir de séquestration de l'agriculture est un enjeu majeur, comme nous le rappelle le programme « 4 pour 1 000 La valeur et l'existence même des paysages ruraux relèvent de la notion de bien commun de la société. Notre comptabilité nationale et celle des autres Européens ne sont pas aujourd'hui adaptées à la prise en compte de ce patrimoine naturel. européenne ouvre cette réflexion indispensable en demandant la création d'une prestation pour service environnemental ou écosystémique qui serait versée aux agriculteurs en fonction de leur contribution aux enjeux de transition pour lesquels la France et tous les autres pays européens ont pris des engagements devant les citoyens du monde. Dans le domaine des accords commerciaux, au-delà de l'absolue nécessité d'une concurrence loyale et équilibrée protégeant nos signes d'identification de la qualité et de l'origine, nous rappelons l'enjeu de préservation des relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Je pense qu'il faudra aussi très vite mesurer les conséquences que pourraient avoir les ruptures profondes que les États-Unis sont en train d'introduire dans les échanges mondiaux. en seront les conséquences pour l'agriculture française et pour les échanges agroalimentaires ? Mes chers collègues, que le budget de la PAC se maintienne ou non, il y a nécessité de rendre souples et agiles les crédits correspondants, qu'ils soient affectés au premier ou au second pilier, La filière viticole a donné l'exemple il y a quelques années en réinterrogeant sa stratégie et son rapport à la PAC. L'exemple n'est peut-être pas transposable à toutes les filières, mais il mérite d'être connu. Vigilance et responsabilité ont guidé les travaux de notre groupe de suivi- cette proposition de résolution européenne en est la parfaite illustration. Nous attendons maintenant, monsieur le ministre, de savoir comment le Gouvernement entend entend préserver les intérêts agricoles et agroalimentaires de la France tout en ouvrant des perspectives nouvelles et réalistes pour soutenir durablement l'ensemble de ses agriculteurs et des territoires concernés. La parole

la première résolution du Sénat, celle du 8 septembre 2017, visait à envoyer « un message politique fort adressé au président de la Commission européenne et au président du Parlement européen qui renforcera utilement les efforts déjà engagés par les pouvoirs publics français pour faire entendre la position française sur l'avenir de la politique agricole commune Il est à craindre que ce message politique très fort n'ait pas ou guère été entendu, d'où l'urgence d'en formuler un second en des termes plus précis. Cette fois, il s'adresse plus encore aux autorités politiques françaises afin qu'elles fassent valoir cette position au Conseil. Dans la foulée des interventions de mes collègues rapporteurs, je souhaite, pour ma part, insister sur deux points. En premier lieu, notre proposition de résolution européenne met l'accent, à dessein, sur ce qui constitue le coeur de la prochaine réforme aux yeux de la Commission européenne, c'est-à-dire le mécanisme de mise en oeuvre de la PAC.

Nos craintes sont partagées par nombre d'observateurs. À titre d'illustration, je citerai ici les propos de Luc Vernet au nom de : « La Commission propose une PAC nationalisée ou régionalisée, moins politique et plus technocratique, où elle garderait un droit de veto systématique. Il ne s'agit en aucune façon d'une simplification. Au surplus, l'expérience des plans de développement régional du second pilier, dont la complexité byzantine est unanimement reconnue, laisse perplexe. Les risques de distorsion de concurrence sont élevés : certains États membres pourraient être tentés d'utiliser le principe de subsidiarité pour gagner en compétitivité grâce au moins-disant réglementaire. Inversement, d'autres pays, dont la France, pourraient vouloir aller au-delà des normes européennes. Monsieur le ministre, est-ce vraiment cela que nous voulons ? J'en arrive, en second lieu, au qui se dessine sur les règles de concurrence et de gestion des crises après les avancées introduites par le « Règlement Omnibus ». La Commission européenne semble s'en satisfaire. Notre proposition de résolution européenne fait valoir que ce règlement ne constitue qu'une étape dans la voie d'une meilleure sécurisation des revenus des agriculteurs. Six autres points sont ensuite consacrés aux progrès souhaités par vos rapporteurs tant en matière de gestion des risques que de modalités d'intervention sur les marchés en période de crise ou d'adaptation des règles de concurrence. Monsieur le ministre, la prochaine réforme de la PAC ne pourra éluder les sujets de la rémunération des agriculteurs, du fonctionnement des marchés et de la volatilité des cours des produits agricoles. À défaut, elle marquerait un renoncement, faute de consensus européen, comme l'a justement souligné le professeur Jean-Christophe Bureau dans un entretien publié avant-hier. En définitive, il semblerait, pour reprendre les mots employés par Paul Verlaine dans son célèbre poème, qu'un vent mauvais souffle sur la prochaine réforme de la PAC.

Il n'est peut-être pas encore trop tard pour inverser le cours des choses. Cela supposerait, en particulier, que les autorités politiques françaises envoient désormais des messages univoques. Très À tort ou à raison, certains de nos partenaires ont manifestement interprété la période récente comme celle d'un de la position suivie par la France depuis 1962. Monsieur le ministre, si notre pays ne défend pas la PAC, qui le fera ? Très bien

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le président de la commission des affaires européennes, messieurs les rapporteurs, madame la rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous y préparions tous depuis de nombreux mois : la Commission européenne a publié, le 2 mai dernier, son projet de budget pour la prochaine période de programmation post-2020 et, le 31 mai, ses projets de règlement de la future politique agricole commune. Nous entrons donc dans une nouvelle phase de discussion et de travail. Dès ma prise de fonction, j'ai organisé de nombreuses réunions sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs concernés. J'ai notamment

La PAC est l'une des plus anciennes politiques européennes- cela a été rappelé. Elle est la seule qui soit véritablement intégrée et, de ce fait, elle est un symbole pour l'ensemble du projet européen. Elle n'est pas parfaite, nous le constatons tous, mais elle a su évoluer au fil des années pour s'adapter. Ce que je retiens de ces échanges, c'est d'abord un impérieux besoin de simplification. Nous avons atteint un niveau critique, et la prochaine réforme de la PAC ne sera réussie que si elle apporte de réelles améliorations, avant tout, pour nos agriculteurs. Cette simplification doit permettre aux agriculteurs de se recentrer sur leur métier, et la nouvelle PAC devra libérer leur capacité à innover, à se moderniser, à fournir non seulement une alimentation de qualité et durable, mais aussi l'énergie ou des matériaux de demain. En résumé, et c'est là l'essentiel, la PAC doit accompagner la transformation de l'agriculture européenne. Nous l'avons vu tout au long des discussions qui se sont tenues dans le cadre des états généraux de l'alimentation, ce sont toutes les filières qui doivent se transformer, être mieux structurées afin de mieux répartir la valeur ajoutée et d'aboutir à des prix raisonnables pour tous. La PAC doit permettre d'accompagner les plans de filières. Elle doit continuer à être une politique tournée vers l'avenir, qui renforce la position des agriculteurs dans les négociations commerciales. Mais tout cela ne sera possible que si les agriculteurs, et au premier chef les nouveaux installés, peuvent se prémunir contre les aléas de tous ordres : les événements climatiques extrêmes, les crises sanitaires et, de façon générale, les aléas économiques et la volatilité des prix. L'agriculture européenne, singulièrement l'agriculture française, est ouverte sur le monde. Nous importons des produits, nous en exportons également Nous pourrions d'ailleurs mieux accompagner nos producteurs pour gagner des parts de marché à l'export ; nous nous devons d'être offensifs en la matière. Mais nous avons également des filières sensibles, stratégiques, que nous devons protéger, soutenir, défendre. Nous sommes dans une phase de négociations commerciales bilatérales intenses. L'Union européenne, après avoir négocié avec le Canada, se prépare à entrer dans une phase finale avec le MERCOSUR et à ouvrir de nouvelles négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. À ce sujet, je porterai un message clair partout où cela sera nécessaire : nous devons nous assurer que les politiques européennes sont cohérentes entre elles. Nous ne pouvons pas soutenir des filières sensibles grâce à la PAC, d'un côté, et ne pas les protéger dans les négociations commerciales internationales, de l'autre. Il serait inacceptable

Nos agricultrices et nos agriculteurs, les femmes et les hommes qui travaillent dans nos secteurs agricoles et agroalimentaires, doivent disposer de toutes les garanties pour faire face à ces aléas. Pour cela, j'attends que les outils de gestion des risques soient au coeur de la future PAC. De ce point de vue, pour moi, cela ne fait absolument aucun doute : les aides directes du premier pilier, découplées et couplées, constituent la première maille du filet de sécurité. Mais la PAC doit aller plus loin, beaucoup plus loin, car les aléas climatiques, notamment, sont nombreux et de plus en plus violents. Nous l'avons vu récemment avec les terribles orages qui se sont abattus sur notre pays et ont partiellement- parfois, totalement -détruit les récoltes à venir. Ces aides doivent également s'accompagner d'une responsabilisation de chaque acteur au sein des filières. Bien sûr, il faut que la PAC prévoie des outils pour que les agriculteurs disposent rapidement et facilement d'une aide de trésorerie. En ce sens, la réserve de crise doit absolument évoluer pour être d'utilisation plus souple. Tous les outils qui permettent d'agir sur le marché doivent être préservés : stockage public et privé, possibilité de réduire volontairement la production, comme cela a été fait lors de la crise laitière en 2016. Tout cela doit être fait plus rapidement, plus efficacement, sans attendre que la situation se dégrade. Nous avons donc besoin d'observatoires des marchés opérationnels et réactifs. Il Il faut aussi que la PAC accompagne les agriculteurs pour faire face aux autres urgences, notamment le changement climatique. L'agriculture fait pleinement partie de la solution pour affronter cette question à travers le stockage du carbone, ... Exactement au développement de nouvelles filières autour de la bioéconomie et de la chimie verte. L'agriculture est le seul secteur capable d'offrir aujourd'hui une alternative crédible à l'utilisation des matériaux fossiles. La PAC doit accompagner l'agriculture dans la mutation de toute notre société vers une économie bas-carbone. De façon plus générale, les préoccupations environnementales doivent être pleinement intégrées à la PAC. Beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les pratiques ; il faut continuer et amplifier ce mouvement. La préoccupation environnementale n'est pas une lubie. Agir en faveur de la biodiversité et participer à l'amélioration de la qualité des eaux, de l'air ou du bien-être animal concourent à faire de l'agriculture européenne celle ayant les plus hauts standards au monde. Nous devons en être fiers et aller encore plus loin, en favorisant tous les dispositifs de qualité, l'agriculture biologique, mais aussi les autres schémas de certification. De ce point de vue, la présence dans la proposition de la Commission européenne d'un instrument en faveur de l'environnement dans le premier pilier de la PAC est une bonne nouvelle. Les propositions de règlement que la Commission européenne a publiées le 1 juin nous permettront-elles de faire tout cela

Cette nouvelle PAC nous permettra-t-elle d'innover, de moderniser les systèmes de production et de défendre nos exploitations familiales dans une économie mondialisée ?

Nous devrons négocier cette politique à vingt-sept avec des logiques parfois totalement différentes. Il faudra prendre en compte non seulement la position des autres membres du Conseil, mais aussi celle du Parlement européen, l'autre colégislateur. Comme je l'indiquais, des choses positives figurent d'ores et déjà dans les projets présentés par la Commission européenne, mais certaines orientations méritent d'être éclaircies. L'un de mes points principaux d'attention concernera les aspects liés à la gouvernance. Nous ne pouvons qu'être satisfaits que la Commission européenne propose une approche stratégique globale, qui soit souple et source de simplification pour les bénéficiaires de cette politique. Cela peut permettre de répondre à notre demande de subsidiarité : les mesures européennes doivent pouvoir s'adapter à nos territoires, si variés en Europe. Ces plans stratégiques, qui doivent décrire la façon dont les États mettent en oeuvre à la fois le premier et le second pilier, permettront d'intégrer des objectifs européens de façon transversale. Ainsi, les questions environnementales doivent être abordées aussi bien à travers le premier pilier, avec la conditionnalité ou la rémunération des services environnementaux, qu'à travers le deuxième pilier, avec les mesures agroenvironnementales et climatiques. Les plans stratégiques doivent permettre de s'assurer que toutes les mesures de la politique sont cohérentes et que les lignes de partage entre les différents dispositifs et la répartition des responsabilités sont claires. Cependant, sous prétexte d'une flexibilité et d'une simplification qui ne concerneraient que la seule Commission européenne, cette démarche ne peut pas et ne doit pas se traduire par un risque de distorsion de concurrence entre les États membres de l'Union. La PAC doit rester, par construction, une politique européenne, et les obligations doivent être les mêmes pour tous les agriculteurs européens. Vous l'aviez souligné dans votre rapport de juillet 2017, toute renationalisation, même partielle, serait un coup fatal porté à cette politique- je partage pleinement cette orientation. Dans les mois à venir,

sur ma combativité, mon énergie et ma mobilisation pour la faire entendre. Cela commence par le nerf de la guerre : le budget. Accompagner cette grande transformation de l'agriculture européenne ne se fera pas sans argent. Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Le 2 mai dernier, la Commission européenne a proposé un budget global pour l'Union européenne à vingt-sept en augmentation, mais, dans ce budget, la PAC est en baisse de 5 % en euros courants, c'est-à-dire sans prendre en compte l'inflation. En réalité, donc, c'est une baisse de plus de 15 %, si l'on prend en compte l'inflation, et elle atteint 25 % pour le second pilier de cette politique. Un quart du budget C'est donc la seule PAC qui participerait au financement du départ du Royaume-Uni ! Pourquoi le revenu des agriculteurs européens devrait-il baisser en raison du départ d'un État membre ? Je l'ai dit dès le premier jour, dit dès le premier jour, et je le redis : c'est inacceptable ! Je consulte l'ensemble de mes partenaires européens. Le 31 mai dernier, avec mes homologues espagnol, portugais, irlandais, finlandais et grec, nous avons créé le groupe de Madrid,

courir le risque de voir la viabilité de leurs exploitations remise en cause. Je compte saisir toutes les opportunités pour défendre l'ambition qui est la nôtre un budget stable pour une PAC renouvelée, simple et efficace. Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis favorable à l'adoption de cette

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

; ils se trouvent aux prises avec la volatilité des marchés mondiaux ; l'agriculture est à la base de notre culture et de notre civilisation ; sans les agriculteurs, notre sécurité alimentaire ne serait plus qu'un leurre. Aujourd'hui, notre vigilance sur les difficultés qu'ils rencontrent est essentielle, elle demeurera constante et indéfectible. Je souhaite aussi remercier mes collègues du groupe de suivi de la PAC pour le travail constructif et transpartisan que nous menons ensemble depuis plusieurs années déjà, en particulier lors de ces derniers mois où les auditions ont été d'une grande richesse. Le projet de budget de la PAC proposé par la Commission européenne est désormais connu et, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, il conduirait à des baisses drastiques et insoutenables de revenu pour nos agriculteurs. Les défis actuels auxquels fait face l'agriculture européenne sont si nombreux qu'il serait incompréhensible qu'une telle réduction budgétaire soit entérinée. Comment, avec une telle baisse du budget, ne pas craindre pour la viabilité de nos exploitations ? Comment accompagner la transition de notre agriculture vers des systèmes plus durables et résilients ? Comment réparer les conséquences encore visibles des crises passées ?

Rappelons que la PAC est la politique la plus intégrée de la construction européenne. Bien que perfectible, elle est l'une des réussites de ce projet européen, mais elle est aussi la pierre angulaire de notre sécurité et de notre souveraineté alimentaires, nationales comme européennes. En effet, dans les négociations commerciales qu'elle mène au nom de ses pays membres, l'Union européenne a fait de la défense de standards élevés de qualité, sanitaires et environnementaux, tout comme de la promotion de ses indicateurs géographiques, un point offensif. Nous approuvons évidemment cette démarche. Ces normes élevées sont une force et font de l'Union européenne l'une des principales puissances agricoles du monde. Or la PAC contribue pleinement à rendre ces standards possibles. De même, elle sera demain l'une de nos réponses aux défis climatiques, qui nous frappent déjà de plein fouet. Soyons donc cohérents et ne défendons pas d'un côté des normes que nous affaiblissons nous-mêmes de l'autre ! Nous en convenons : la PAC doit être modernisée. Elle souffre d'imperfections et de complexités, qui l'empêchent d'être pleinement efficace. Toutefois, nous refusons que cet effort de simplification se fasse au détriment de l'essence même de ce qui la caractérise : incarner une politique commune qui protège les agriculteurs comme les consommateurs. Il n'est pas question de sacrifier ce trait de caractère de la PAC, et je dirais même ce trait de valeur, qui a été si ardemment défendu. Les objectifs poursuivis par ce projet de réforme de la Commission européenne sont louables sur le papier. On ne peut qu'y souscrire. Je pense par exemple à la simplification visant à atteindre une meilleure efficacité, à l'établissement d'une allocation plus juste des aides directes, aux ambitions plus élevées en matière d'environnement et d'action pour le climat ou à l'attention portée aux jeunes dans un contexte où seuls 6 % des agriculteurs européens ont moins de trente-cinq ans. Cependant, des interrogations subsistent. Parce que le temps me manquera, je ne partagerai avec vous qu'une seule de mes réflexions ; elle concerne les plans stratégiques nationaux agricoles.

Cette crainte est légitime, dès lors que les conditions d'attribution des aides ne seront plus identiques pour l'ensemble des États de l'Union européenne et qu'elles seront seulement guidées par des principes généraux. Certains États pourraient être tentés d'utiliser le principe de subsidiarité pour gagner en compétitivité, en ayant recours au moins-disant réglementaire. Inversement, d'autres pays, dont le nôtre, pourraient vouloir aller au-delà des normes minimales européennes. Même si le commissaire Phil Hogan tente de nous rassurer et nous promet que la Commission européenne veillera à éviter de telles distorsions, ces scénarios ne sont pas fantaisistes, puisqu'ils se réalisent sur d'autres sujets.

la négociation du prochain cadre financier européen pour la période 2021-2027 aurait pu être l'occasion de recadrer, réorienter, la politique agricole commune, mais, encore une fois, l'occasion est manquée.

les nouvelles priorités politiques de l'Union européenne. Si le financement de ces priorités est nécessaire, cela ne doit pas se faire au détriment de l'agriculture. Nous soutenons donc la démarche de nos collègues, en particulier sur la nécessité d'une adaptation du droit de la concurrence au secteur agricole, d'un renforcement du poids des producteurs dans la chaîne alimentaire ou encore d'un renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales des firmes transnationales et contre les pratiques des centrales d'optimisation fiscale du secteur de la distribution.

Ce faisant, elle bénéficie principalement aux gros producteurs. L'objectif d'accroissement de la productivité a pris le pas sur les autres objectifs et a provoqué la disparition massive des petites exploitations jugées moins rentables et moins capables de faire face aux défis de la concurrence, cadre de l'OMC, qui exige que l'Union européenne aligne ses prix agricoles sur les cours mondiaux. Il y a donc ceux qui s'enrichissent- 84 % des aides vont à 20 % des agriculteurs -et les petits exploitants qui ne s'en sortent pas. La tentative

Il est urgent que l'Europe mette en place une nouvelle politique agricole commune, intégrant un véritable plan stratégique de souveraineté et de sécurité alimentaires, et qu'elle cesse de sacrifier son agriculture sur l'autel du libre-échange. que cessent les concessions agricoles accordées dans les négociations commerciales- MERCOSUR, CETA, etc. -, qui menacent des pans entiers de l'agriculture européenne et nombre de nos territoires. De plus, pour nous, comme pour nos collègues députés européens, il faut sortir la PAC de cette politique productiviste mortifère. Entre le flux des paiements indiscriminés du premier pilier, dont une proportion échappe aux aux agriculteurs et dont les effets redistributifs posent question, et l'éparpillement du second pilier entre des objectifs très variés, la politique agricole commune n'a plus de véritable orientation. À l'inverse, nous voulons une agriculture familiale, locale, permettant une production de qualité, un « réinvestissement » des campagnes et une transition écologique et ayant pour objectifs la souveraineté alimentaire et une rémunération juste pour celles et ceux qui travaillent la terre. la terre. Pour cela, nous demandons une relocalisation de la production afin de favoriser les circuits courts, qui permettent une meilleure traçabilité des produits et favorisent de nouvelles formes de distribution. une redirection des aides vers les exploitations paysannes en faveur de la transition écologique ; une sortie du glyphosate et des substances nocives pour la santé et l'environnement, tout en accompagnant financièrement les agriculteurs une production axée sur la transition écologique, en favorisant la rotation des cultures et en refusant les OGM ; la mise en place des réformes foncières par les États membres pour lutter contre la spéculation sur les terres et l'étalement urbain des instruments publics de régulation de la production- réinstauration de quotas pour sortir de la logique de surproduction, maintien des droits de plantation des vignes la mise en place d'un système européen de garantie de la propriété publique du patrimoine génétique animal et végétal pour éviter son appropriation par les multinationales ; la mise en place d'agences publiques de certification et de contrôles des productions bio et des labels afin de favoriser les savoir-faire

toutes les informations qui nous parviennent sur la réforme de la PAC nous alarment, pour trois raisons. D'abord, la réforme de la PAC s'inscrit dans un contexte complexe : celui de l'élaboration du prochain cadre financier marqué, d'une part, par les conséquences financières du retrait britannique et, d'autre part, par les nouveaux défis posés à l'Europe, qui se traduiront par de nouvelles priorités politiques et budgétaires. Ensuite, des réductions drastiques sont annoncées. Enfin, l'agriculture européenne, notamment française, est fragilisée par les crises des dernières années. Nos agriculteurs, dont un tiers perçoivent 350 euros par mois, vivent des situations dramatiques. Dans ce contexte, et au vu des éléments préparatoires de la Commission européenne, le signal d'alarme que constitue cette proposition de résolution européenne est plus que nécessaire. J'en salue les auteurs et rapporteurs, qui lancent un appel clair au niveau institutionnel français, ainsi qu'au plan européen. Si nous voulons conserver notre statut de première puissance agricole mondiale et renforcer le poids de nos secteurs agroalimentaires, un budget stable et ambitieux s'impose.

et de sauvegarder une politique historique, symbole de l'ambition européenne. Ainsi donc, il s'agit aujourd'hui de se poser les bonnes questions et de retrouver le sel. La PAC n'est pas seulement une affaire budgétaire : c'est la colonne vertébrale de notre modèle agricole. Quelle alimentation voulons-nous réellement en Europe ? Quelle agriculture pour nourrir sainement 500 millions de consommateurs européens ? Quelle agriculture pour peupler nos territoires et les rendre dynamiques et attractifs ? Quelle durabilité de notre modèle agricole ? Quelles relations commerciales pour défendre nos intérêts ? Comment poursuivre le défi de l'autosuffisance alimentaire à l'échelle de notre continent ?

pleinement. Par ailleurs, je tiens à souligner que le redécoupage des zones défavorisées tel qu'il a été acté est une hérésie sur certains territoires de France et qu'il s'opérera au détriment de la préservation de l'emploi et de la diversité des territoires. Nombre d'exploitants exclus de la future carte attendent, monsieur le ministre, des réponses de votre part. Le sentiment d'abandon est très présent dans l'agriculture française. Nous formons donc le voeu que les négociations à venir et le budget européen aboutissent dans un sens qui dote l'Europe des moyens nécessaires à une ambition franche pour notre agriculture européenne. Cela passe aussi par la question des ressources budgétaires de l'Union européenne. À cet égard, monsieur le ministre, qu'en est-il de la position du Gouvernement au sujet de l'augmentation du budget européen et des ressources propres ? La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier personnellement M. Daniel Gremillet, Mme Pascale Gruny et MM. Claude Haut et Franck Montaugé, auteurs de cette proposition de résolution européenne « en faveur d'une Politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires À la veille des débats sur le projet de loi portant sur l'agriculture et l'alimentation, cette proposition de résolution européenne tient lieu de signal d'alarme. Dans ses propositions relatives au cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission européenne propose une réduction de 5 % du budget de la politique agricole commune en euros courants. Les aides directes aux agriculteurs, qui représentent pourtant une part non négligeable des revenus de ceux-ci, accuseraient une baisse de 4 % en euros constants, soit 80 % de la baisse annoncée du budget total. En opérant une coupe budgétaire drastique, cette proposition de la Commission européenne revient à faire de la politique agricole commune une variable d'ajustement du budget européen et à considérer l'agriculture comme une simple valeur ajoutée à l'architecture européenne, alors qu'elle en est le ciment. En réaction à cette offensive, la présente proposition de résolution européenne vise à garantir des ressources budgétaires stables et suffisantes pour soutenir les producteurs et encourager l'évolution de notre modèle agricole. Nous attendons notamment une évolution du droit de la concurrence. Il est urgent que le droit européen s'adapte aux spécificités du monde agricole. À cet égard, j'ai présenté en commission des affaires économiques un amendement visant à formaliser une demande de reconnaissance des circuits de proximité. Dans le droit européen, en effet, les règles des marchés publics sont contraignantes et ne permettent pas de privilégier l'approvisionnement dit de proximité en produits locaux, par exemple pour alimenter la restauration scolaire. La libre La libre concurrence ne doit pas se faire au détriment de nos territoires ! Nous devons ouvrir notre commerce à l'extérieur, sans perdre le lien local. Cet amendement, cosigné par plus de quarante de nos collègues, exprime d'abord une volonté qui émane de nos élus locaux. Ainsi, dans le Nord, des maires mènent une résistance exemplaire pour permettre aux enfants de leur commune de manger sainement, avec des produits frais issus des exploitations voisines. La demande est forte en matière de circuits de proximité. Pour autant, je ne saurais recommander à l'agriculture française de se replier sur elle-même. Je plaide pour un développement agricole équilibré si des secteurs tels que les produits maraîchers et la viande se prêtent aux circuits courts, il en va autrement pour les secteurs d'exportation que sont les céréales, le vin, l'huile de colza ou encore la pomme de terre. N'oublions pas les circuits longs ! Une bouteille sur dix de vin français est consommée en Chine et 90 % des productions de cognac sont exportées Or la volonté de réduire le budget de la politique agricole commune entre en contradiction avec les choix géostratégiques opérés par les autres grandes puissances agricoles mondiales, à commencer par la Chine, les États-Unis et la Russie. « L'agriculture est la locomotive de l'économie russe », a dit Vladimir Poutine. Ne laissons surtout pas à la Russie le monopole de la diplomatie agricole ! La France est douée pour négocier des Airbus, des Rafale, mais quelle est sa stratégie en matière d'exportations agricoles ?

en 2050, les besoins en céréales auront décuplé sous les effets du changement climatique, de la croissance démographique et des flux migratoires. Diminuer les aides de la politique agricole commune, c'est oublier que la surproduction nationale bénéficie à des millions de personnes vivant hors de nos frontières ; c'est oublier aussi que ces exportations participent à la balance commerciale de la France. L'Europe est avant tout une puissance agricole : ne sacrifions pas le budget de la politique agricole commune sur l'autel des nouvelles priorités européennes

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite que notre assemblée se penche cet après-midi sur l'avenir et le budget de la politique agricole commune. Le sujet est d'une actualité brûlante, puisque, vendredi dernier, la Commission européenne a dévoilé ses propositions, non sans susciter de vives inquiétudes. Les eurodéputés ont manifesté de fortes réserves, qu'ils ont formalisées dans une résolution adoptée à une large majorité. C'est un signal qui rejoint, monsieur Gremillet, celui

En effet, ils n'ont pas manqué de tirer la sonnette d'alarme. Oui, pour ne pas les citer, la PAC pourrait « traverser un cap dangereux en 2020 On le sait, en l'état des négociations, si rien n'est fait, la PAC pourrait être une variable d'ajustement des conséquences budgétaires du Brexit- de 10 milliards à 13 milliards d'euros en moins -et de l'émergence de nouvelles priorités politiques, notamment en matière de sécurité, de migration et de défense.

Alors que cette politique fondatrice de l'Union européenne est garante de la sécurité et de l'autonomie alimentaires de celle-ci, elle ne pèserait plus que 28,5 % au sein du budget de l'Union européenne, contre 37 % aujourd'hui. Il serait tout à fait paradoxal que l'Europe se désarme dans ce domaine, au moment où, au contraire, les grandes puissances économiques telles que le Brésil, l'Inde, la Russie ou les États-Unis investissent lourdement dans leur indépendance alimentaire, donc dans leur politique agricole. Nous ne pouvons accepter cette baisse drastique, et vous avez dit à plusieurs reprises, monsieur le ministre, que vous ne l'acceptiez pas non plus. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé et compte tenu des différents aléas auxquels doit faire face notre agriculture, une politique européenne de soutien demeure essentielle à la viabilité de nombreuses exploitations agricoles en France. En effet, les aides représentent aujourd'hui en moyenne 47 % du revenu des agriculteurs français. Une perte de 5 milliards d'euros d'aides directes au cours de la période 2021-2027 est donc inenvisageable pour notre pays. Certes, l'Europe peut porter une ambition agricole commune rénovée et encore mieux adaptée aux nouvelles exigences économiques, environnementales et de consommation. Les agriculteurs se sont toujours montrés ouverts à la modernisation, pourvu qu'elle soit porteuse de sens et source de simplification. En conséquence, sur les grandes lignes, on doit pouvoir obtenir un consensus au sein de l'Union européenne pour l'accompagnement des exploitations dans leur développement et leurs innovations, la gestion et la prise en compte des changements climatiques, l'aide à la modernisation des entreprises, l'appui à la structuration de filières modernes pour mieux organiser la production production et, surtout, la fondation d'une politique véritablement commune de gestion des risques agricoles et de gestion de crise. Je regrette que la Commission européenne manque particulièrement de volontarisme sur ce point. tout cela sera difficile à réaliser si la PAC n'est pas maintenue dans une dynamique budgétaire. Au-delà des considérations financières, la Commission européenne propose une méthode de mise en oeuvre de la PAC qui risque de poser problème. Les organisations agricoles se sont inquiétées, à juste titre, du principe de subsidiarité, qui entraînerait des distorsions de concurrence entre les agriculteurs européens, ce que la PAC est pourtant censée éviter. Même si les plans stratégiques des États membres seront soumis à un contrôle, ne s'oriente-t-on pas vers une renationalisation rampante des aides ? Au RDSE, nous sommes fermement opposés à toute forme de renationalisation de la PAC en ce qui concerne le premier pilier ! Je n'oublie pas non plus la pression exercée pour harmoniser les montants des paiements directs. Pour autant, il ne s'agit pas de s'enfermer dans un conservatisme ; mais garantissons une politique commune avec un grand « C » ! Pour cela, maintenons un socle de règles standards et de soutiens financiers communs, qu'une politique de marché, tout en garantissant à chaque État une marge de manoeuvre raisonnable et réaliste. S'agissant du second pilier, conçu comme porteur d'une politique territoriale, voire territorialisée,

L'agriculture européenne a besoin aussi d'un soutien modernisé, à travers la mise en place de nouveaux outils. Je pense en particulier au statut de l'agriculteur, qui doit avancer afin de permettre une meilleure répartition des aides.

Il faut notamment renforcer les mécanismes assurantiels et de gestion de crise pour pouvoir soutenir la résilience des exploitations agricoles face à la volatilité des prix et aux aléas climatiques. La présente proposition de résolution européenne le suggère. Il faut aussi réaffirmer une politique ambitieuse en matière de diversité des cultures, notamment en direction des cultures sources de protéines, des légumineuses et des protéagineux. Il me paraît également important de soutenir et de sécuriser les filières d'agrocarburants, afin de rendre l'Europe moins dépendante des énergies fossiles. Elles Elles sont aussi une source importante de protéines. Mes chers collègues, le Sénat a toujours été très attentif à l'avenir de la PAC, sans pour autant ignorer l'intérêt des autres politiques européennes, ô combien nécessaires. Le RDSE, très attaché à l'Europe, est soucieux de l'équilibre à trouver sur le plan budgétaire pour faire coexister toutes les priorités et toutes les attentes de nos concitoyens. Seul un budget à la hauteur des défis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution européenne revêt un caractère extrêmement important, puisque, entre les défis actuels et futurs pour notre agriculture et les annonces de la Commission européenne, un fossé abyssal est en train de se creuser. Si nous partons du postulat, fort probable, que la population mondiale atteindra 9 milliards d'habitants en 2050, la sécurité alimentaire est une problématique cruciale. Peu de pays au monde ont la chance d'avoir un climat tempéré et permettant une production agricole sereine. La France a cette chance, doublée par le fabuleux avantage de la multiplicité de ses territoires, qui contribue à offrir un panel de produits exceptionnels. L'agriculture a aussi le fabuleux pouvoir de façonner les paysages partout dans le pays, faisant l'ébahissement de millions de touristes. Cela a été jusqu'à présent possible, car nous avons toujours favorisé le maintien d'une agriculture familiale, répartie dans toutes les régions de France. C'est aussi le fruit d'une politique sachant corriger les écarts : la compensation des handicaps naturels, à travers notamment l'ICHN, a été un des éléments les plus aboutis d'une prise en compte des différences de productivité entre la plaine et la montagne. Tous ces éléments devraient nous permettre de croire à un avenir meilleur pour l'agriculture française : elle aurait un rôle central dans le défi de nourrir le monde et éviterait que des millions de personnes soient réduites à quitter leur pays et à migrer à la recherche hypothétique d'une vie meilleure. Eh bien non, monsieur le ministre, rien de ce que l'on entend ou lit aujourd'hui des communiqués de la Commission européenne ne nous permet de croire à un avenir meilleur pour nos agriculteurs En effet, l'annonce de la diminution de 5 % du budget de la PAC nous fait froid dans le dos, d'autant plus que ce chiffre cache une réalité encore plus sombre : une baisse réelle de 14,7 % sur le premier pilier et de 26,3 % sur le second. Vendredi dernier, la Commission européenne a même annoncé le passage des cofinancements obligatoires des États membres pour le second pilier de 25 % à 57 %, ce qui engendrera une dépense supplémentaire pour l'État français de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

En cherchant bien, je trouve des éléments de réponse, dont le premier se trouve dans le discours prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne, le 26 septembre dernier. Le Président de la République a insisté pour ouvrir un débat décomplexé sur la PAC, en en critiquant d'ailleurs les contours, tout en proposant de nouvelles politiques européennes, comme la défense Comment n'avoir pas compris que, dans une Europe déchirée par le Brexit, avec la situation instable de pays comme l'Italie ou l'Espagne et des pays de l'Est qui ne voient dans la PAC qu'une source de financement social de leurs populations rurales, le risque d'ouvrir la boîte de Pandore était réel ? Et que le résultat de ces annonces ne pouvait que faire baisser le premier budget européen que constitue la PAC ? Comment ne pas comprendre, quand on est Président de la République française, que, lorsqu'on demande de faire plus à l'Europe, alors que, dans le même temps, nous ne le pouvons pas, asphyxiés que nous sommes par nos dépenses publiques et notre dette, cela ne peut qu'accélérer une diminution du budget de la PAC De plus, dans ce même discours, Emmanuel Macron a proposé plus de subsidiarité des États membres dans l'application des modalités de la PAC. Cela me fait craindre le pire et m'amène à ma deuxième réponse.

cesse entre une agriculture économiquement productive et une agriculture qui se plierait au diktat de l'écologie punitive, passéiste, recroquevillée sur elle-même, où tout passe

Ce manque de cap de nos ministres successifs, qui a contribué à rendre la voix de la France dans le domaine agricole inaudible, laisse la plus grande place à nos concurrents Nord-européens, qui, eux, ont bien compris que l'agriculture est un formidable levier de croissance et de création de valeur, tant sur le marché intérieur qu'à l'export. Alors, monsieur le ministre, il faut vous ressaisir fort la voix de la France agricole ! Ne restez pas en retrait des discussions européennes ! Gambetta, en 1883, avait voulu faire chausser les sabots de la République aux paysans ; cela a été une réussite, tant les agriculteurs ont contribué à l'effort pour faire une France solide. Ne les décevez pas, ne les déchaussez pas : ayez le courage d'affirmer que la France est un grand pays agricole et que l'agriculture française est largement capable de relever le défi de nourrir les Français et bien d'autres

On fait dire aux chiffres ce que l'on veut. Aujourd'hui, nous savons que la Commission européenne propose une baisse de 5 % de la PAC : 365 milliards d'euros

L'annonce de la diminution du budget français de la prochaine PAC a produit ses réactions immédiates : un mélange d'indignation et de colère, avant le désespoir. Mais il ne suffit pas de dire que les propositions de la Commission européenne sont inacceptables ; il faut agir Mes chers collègues, si nous voulons être honnêtes, nous devons admettre que cette annonce n'est pas une surprise. En effet, face aux autres enjeux de l'Europe- Brexit, gestion de la politique migratoire, de la défense et du numérique -, nous savions que la PAC serait menacée. Quelles que soient nos convictions politiques, nous devons reconnaître à Stéphane Le Foll la ténacité avec laquelle il a arraché, à la force des poignets, le maintien du budget précédent. Nous savions que, pour la nouvelle PAC, ce serait encore plus difficile. Je vous souhaite, monsieur le ministre, la même réussite. Nous avons été nombreux à affirmer qu'une réforme de la PAC devait intervenir. Appréhender les mutations internationales pour repenser une agriculture au sein de l'Union européenne, c'est d'abord réfléchir aux défis que nous devons collectivement relever maintenir une indépendance alimentaire et la qualité de nos productions, garantir le revenu des agriculteurs en limitant la volatilité des prix, préserver l'environnement et s'adapter aux changements climatiques, répondre aux obligations de sécurité alimentaire et préconiser l'accès à des outils de gestion des risques. Pour cela, il faut une PAC plus équitable. Cela concerne un meilleur ciblage des aides directes sur la diversité des systèmes agricoles, sur les petites exploitations et vers les jeunes, un paiement redistributif obligatoire accordant une aide plus élevée sur les premiers hectares, un plafonnement obligatoire tenant compte de la capacité des exploitations à garder de l'emploi, un paiement à de véritables agriculteurs actifs des paiements assis sur une forte conditionnalité. En juin dernier, je formulais ainsi la problématique : alors que nous nous trouverons en 2017 à mi-parcours, nous devons nous questionner sur ce que la PAC peut encore apporter à l'agriculture française. Comment doit-elle se redéfinir afin de continuer à remplir ses objectifs : assurer un niveau de vie équitable à nos agriculteurs, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables aux consommateurs ? Un an plus tard, les mêmes questions restent posées ... Il n'y a plus de temps à perdre, car, parallèlement à cette annonce de réduction de la PAC, les crises se succèdent, sanitaires, climatiques et économiques, emportant avec elles de nombreux agriculteurs et limitant l'envie des plus jeunes de s'installer. Alors, que faire ? Premièrement, une réorientation en profondeur s'impose. Si la Commission européenne a avancé la grande idée d'un, c'est-à-dire d'un transfert de la gestion de toutes les aides de la PAC aux États membres, cette renationalisation me semble contraire à l'idée même de l'Europe, fondée sur la solidarité et l'interdépendance, avec des objectifs communs pour une agriculture européenne forte.

Les nouvelles orientations vont aggraver cet état de fait. Le rapport Dorfmann sur le futur de l'agriculture et de l'alimentation, réalisé dans le cadre de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen, souligne la nécessité de revenir à la genèse les pays membres doivent suivre un cadre commun de règles européennes très solides, comprenant objectifs, règles de base, instrument d'intervention, indicateurs de contrôle et contributions financières, ce qui éviterait toute distorsion de concurrence.

Il invite aussi la Commission européenne à réaliser des contrôles financiers et de performance et des audits pour s'assurer que le nouveau modèle s'appliquera selon des règles et critères identiques dans tous les États membres. Enfin, dernière mise en garde : ce nouveau modèle de gestion des aides devra respecter l'organisation des pouvoirs de chaque État membre, souvent définie par une constitution. À cet instant, je voudrais souligner l'efficacité et la performance de l'organisation commune du marché vitivinicole, qui a permis d'avoir une viticulture moderne, de restructurer notre vignoble pour correspondre à une demande de qualité et de responsabiliser la filière sur ses choix stratégiques, qui ont montré, depuis sa création, leur efficience.

Une participation jusqu'à 1,3 % du PIB par pays membre, soit une augmentation de 0,2 point de PIB, permettrait tout simplement de maintenir le budget de la PAC en ayant les moyens d'assumer d'autres politiques. du groupe de suivi de la PAC, nous avons reçu au Sénat les attachés des ambassades de plusieurs pays membres : l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie.

Cette nouvelle PAC est primordiale, au-delà même de l'agriculture : le rapport Dorfmann met bien en exergue l'importance du développement rural pour le développement des territoires, la durabilité et l'emploi. Il souligne tout l'intérêt de l'initiative LEADER et des démarches collectives pour valoriser l'ensemble des ressources locales en biens alimentaires, non alimentaires- bioéconomie, énergies renouvelables -et en services, ainsi que pour promouvoir l'économie circulaire. Il insiste aussi sur le maintien des compensations pour les exploitations situées en zone défavorisée. Il propose de créer un nouveau fonds pour les communautés locales de développement, à l'aide d'une réserve de 10 % de tous les fonds structurels. Nous devons collectivement avoir le courage de fixer nos ambitions face aux nombreux défis et nous donner les moyens de réaliser ces ambitions, comme l'ont souligné nos rapporteurs. Monsieur le ministre, sur 100 euros gagnés, un citoyen européen reverse en moyenne 50 euros en impôts et cotisations, dont seulement 1 euro sert à financer le budget de l'Union européenne ... Ainsi, 49 euros restent dans les capitales des États membres. Les pistes existent

Cette politique, qui affecte le quotidien des agriculteurs français, joue un rôle stratégique éminent, notamment pour notre autonomie alimentaire, en France et en Europe. Nous, qui n'avons jamais connu la faim sur notre territoire, ne devons pas oublier l'importance de cette autonomie. Aujourd'hui, monsieur le ministre, alors que cette PAC est en danger, nous regardons ailleurs. Nous nous apprêtons à examiner, d'ici à la semaine prochaine en commission des affaires économiques, et à la fin du mois de juin en séance publique, le projet de loi issu des états généraux de l'alimentation. Ce texte important, qui a bénéficié d'une grande communication gouvernementale, dont je ne vous fais pas grief, monsieur le ministre, met en place des mécanismes pour- encore hypothétiquement -assurer une meilleure rémunération aux agriculteurs. C'est une légitime priorité gouvernementale. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous, en même temps », admettre une réduction directe, brutale et certaine du revenu des agriculteurs par ces coupes claires dans le budget de la PAC ? Les états généraux de l'agriculture ne serviront à rien si la PAC n'est pas au rendez-vous. Pendant que le Gouvernement réfléchissait durant de longs mois, la Commission a rendu ses propositions pour, d'une part, réformer la PAC et, d'autre part, fixer le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Sur les deux tableaux, la France est perdante. Force est de constater

Si nous en sommes là, c'est que la France a été trop absente des réflexions en amont. Ce gouvernement et le précédent ont leur part de responsabilité : si la France avait tenu une position ferme dès le début des réflexions, nous n'en serions pas là. Que penser des paroles du Président de la République à la Sorbonne, en septembre 2017 ? Pour lui, « la PAC est devenue un tabou français ». Il souhaite « que chaque pays puisse accompagner cette transformation selon ses ambitions et ses préférences Quelles sont ces ambitions et ces préférences gouvernementales ? Un budget de la PAC en baisse de plus de 12 % ? Une chute des aides directes, pourtant essentielles dans les comptes d'exploitation de nos agriculteurs Une renationalisation partielle d'une des politiques les plus intégrées de l'Union européenne ? Cette ambition pour la PAC est un changement historique de la position française. Les annonces du commissaire Phil Hogan, la semaine dernière, ont confirmé par ailleurs nos inquiétudes. En permettant à chaque État membre d'adopter un plan stratégique pour atteindre neuf objectifs européens et de disposer de marges de manoeuvre dans l'affectation des dotations, la PAC est indiscutablement en voie de renationalisation. Le risque majeur de cette subsidiarité accrue est évident : creuser encore les distorsions de concurrence entre agriculteurs européens, qui pénalisent déjà en grande partie les agriculteurs français dans de nombreuses filières. Les aides directes sont les grandes perdantes de la réforme proposée, puisqu'elles seront plafonnées. Il convient toutefois de ne pas opposer grandes et petites exploitations, circuits courts et marchés internationaux : la France doit être compétitive sur les deux volets. Surtout, certains points attendus sont totalement absents. Il est notamment inacceptable qu'aucun outil pertinent de gestion des crises ne soit au coeur de la proposition de la Commission dans le contexte actuel de volatilité des marchés. souviens pourtant des engagements du candidat Macron au congrès de la FNSEA, à Brest, en 2017. La position de la France se doit d'être claire : en l'état, elle ne peut accepter de telles orientations. J'ai pris acte de votre volonté d'aller dans ce sens, monsieur le ministre. L'accusation, je le sais bien, est un peu lourde,

Toutefois, monsieur le ministre, cette faute n'est pas inéluctable. Elle peut être réparée. Le temps est compté. Nous avons entendu votre position. Il est grand votre groupe de Madrid, car il est bien tard. Mes chers collègues, la présente proposition de résolution européenne est le fruit d'un travail de plusieurs mois effectué avec talent et obstination par quatre rapporteurs de tous bords politiques. Elle a été adoptée à l'unanimité par la commission des affaires européennes et la commission des affaires économiques,

réalistes, essentielles pour l'avenir de notre agriculture. Son pragmatisme oblige le Gouvernement. Monsieur le ministre, si cette proposition de résolution européenne était adoptée, nous vous engageons à faire valoir cette position au Conseil. Le monde agricole vous observe. Sachez que nous nous tenons à votre disposition pour vous soutenir dans cette démarche.

Il possède quelques dizaines d'hectares de terres. En complément, il fait du maraîchage et de l'élevage pour joindre les deux bouts. Jacques gagne en moyenne 800 euros par mois en travaillant 12 à 15 heures par jour. Sans la PAC, il ne s'en sortirait pas : trop de charges pour trop peu de revenus. La semaine dernière, Jacques m'a interpellé en me disant que les annonces de Bruxelles en vue de la renégociation de la PAC étaient pour lui une véritable catastrophe. Que lui répondre au moment où la Commission européenne avance une baisse drastique de la PAC d'environ 12 %, en tenant compte de l'inflation ? Inacceptable ! Tout simplement inacceptable- je reprends vos propres mots, monsieur le ministre ! « Inacceptable », en effet, si je parle au nom de Jacques et de tous nos agriculteurs et éleveurs français. Aujourd'hui, un nouveau modèle de mise en oeuvre de la PAC, élaboré par la Commission européenne, plaide pour une plus grande liberté laissée aux États. Ce nouveau modèle est en réalité synonyme de distorsion de concurrence et de risque pour le maintien de la qualité des produits. Officiellement, Bruxelles souhaite rendre la PAC plus flexible en laissant les États libres de gérer eux-mêmes une partie des fonds agricoles. Or cette flexibilité ressemble plutôt à un désengagement progressif un désengagement progressif qui aura des conséquences tout à fait dramatiques pour le revenu de nos agriculteurs, déjà en grande difficulté. Que cherche la Commission à travers cette remise en cause de l'esprit et du budget de la PAC ? Tout simplement à se déresponsabiliser et à décentraliser son action. Ce n'est pourtant ni la philosophie de l'Union européenne ni le sens de l'histoire. La PAC, seule compétence pilotée à 100 % par l'Union européenne, est une politique historique, et même constitutive, de l'Europe. La remettre en cause, c'est attenter à l'esprit communautaire imaginé par les pères fondateurs. La PAC est une belle réussite européenne. Elle a permis à des milliers d'agriculteurs d'atténuer le choc de l'exode rural, de l'évolution des modes de consommation et de la mondialisation. Cette PAC a su évoluer en ajoutant au premier pilier, principalement consacré aux aides agricoles, un second pilier dédié au développement rural. En outre, les mesures aujourd'hui avancées par Bruxelles renforcent encore l'inflation administrative, puisque chaque pays, pour soutenir les demandes d'aides, devra présenter un plan stratégique sur la PAC validé par la Commission dans les huit mois, au regard de neuf critères. C'est de cette Europe que ne veulent plus les Européens. C'est de cette Europe que se nourrissent les populismes. Chaque jour, nos agriculteurs et éleveurs français se battent pour imposer un modèle basé sur la qualité, sur le respect des consommateurs et sur la défense d'un savoir-faire agricole. L'Europe leur a donné jusqu'à présent les moyens de tenir ces objectifs et de continuer de vivre dignement de leur travail. Alors que nous attendions de la PAC 2021-2027 des solutions concrètes pour garantir une meilleure rémunération à nos agriculteurs, c'est le contraire qui se produit à travers le renoncement à une politique commune et la baisse très nette du budget de la PAC. En face d'un objectif louable, à savoir une meilleure allocation des revenus agricoles, Bruxelles ne met aucun moyen ni solution adaptés. Les nouvelles priorités de la Commission européenne, à savoir la sécurité, l'immigration et l'environnement ne doivent pas être menées au détriment de l'agriculture. Il y va de la survie de centaines de milliers d'agriculteurs. Il y va de notre modèle agricole. Il y va de la qualité de nos productions. Il y va, enfin, de l'esprit européen. Soyez certain, monsieur le ministre, que nous soutiendrons toute action gouvernementale s'opposant à ce coup de rabot sans précédent et à des mesures dont l'esprit nous paraît si éloigné de l'idéal européen. Nos agriculteurs attendent de nous courage et fermeté pour les défendre. Soyons au rendez-vous de ce combat pour la protection de notre modèle agricole. Aussi, nous soutenons sans réserve la proposition de résolution européenne visant à préserver une politique agricole commune forte et ambitieuse, au service de nos agriculteurs. La parole est à Mme Gisèle

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes très chers collègues, depuis sa création, en 1976, l'indemnité compensatoire de handicaps naturels joue un rôle prépondérant dans le développement rural et le maintien de l'activité économique.

La réforme du zonage en cours de négociation avec la Commission européenne est un sujet d'inquiétude majeur pour nos territoires, nos agriculteurs et nos éleveurs : si elle entraîne des entrées de communes, elle implique 1 341 sorties sur un fondement totalement incompréhensible. Rien n'est Rien n'est prévu pour intégrer les communes exclues de la révision des cartes des zones défavorisées « simples » dans le zonage complémentaire des zones soumises à contraintes spécifiques. De lui-même, ce sujet s'imposait. Le 17 mai dernier, la commission des affaires européennes du Sénat, présidée par M. Jean Bizet, dans toutes ses composantes politiques, a unanimement adopté une proposition de résolution européenne dont je suis l'autrice et que j'ai présentée avec mon collègue Michel Raison.

Ces risques implacables dans toutes les zones concernées sont prégnants en région Occitanie, tout particulièrement dans les départements de l'Aude et du Gers. Derrière un point sur la carte se dessinent de véritables drames humains. Oui, la carte présentée le 20 février dernier est profondément injuste ! Se limiter à des négociations avec la Commission européenne sur des paramètres techniques de l'ICHN condamne à l'impuissance. Il faut donc envisager une approche plus ambitieuse en révisant le coeur du dispositif juridique, c'est-à-dire les articles 31 et 32 du règlement européen du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural. Notre première requête consiste à demander la modification des termes de l'article 31 concernant les critères d'éligibilité des zones soumises à contraintes naturelles et à ajouter des critères obligatoires aux huit critères biophysiques existants.

pour la définition du périmètre des zones soumises à contraintes spécifiques intégrant, de ce fait, des territoires plus étendus, et non uniquement des communes isolées, dans le zonage à contraintes spécifiques, qui se trouvaient jusqu'ici exclus de la cartographie des zones défavorisées simples. convaincue que des outils existent pour réintégrer ces communes et pour les accompagner, je vais vous remettre ce texte afin d'avoir la certitude que le Gouvernement en prenne connaissance et qu'il assume les responsabilités attendues sur ce sujet primordial.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons cette proposition de résolution au moment où le débat sur la PAC après 2020 entre à Bruxelles dans sa phase concrète. Disons-le d'emblée, ce débat s'engage sur des bases extrêmement inquiétantes, notamment au niveau budgétaire. Avec une proposition de 325 milliards d'euros en prix constants, le projet de cadre financier pluriannuel 2021-2027 marque en effet une rupture inédite en matière de budget agricole. Car, si sa part dans le budget général baisse régulièrement depuis trente ans, c'est la première fois qu'il est proposé des coupes claires aussi importantes dans les crédits destinés à nos agriculteurs. Soulignons tout d'abord qu'il s'agit d'un véritable non-sens. Aujourd'hui comme hier, l'agriculture reste une activité éminemment stratégique. Elle le sera sans doute encore davantage demain : l'augmentation de la population mondiale, conjuguée aux dérèglements climatiques et à la pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles, le défi alimentaire au coeur des enjeux fondamentaux du XXIsiècle. États-Unis, Chine, Russie, Inde ou Brésil ne s'y sont pas trompés : depuis une dizaine d'années, les grands pays ont renouvelé leur vision stratégique et n'ont pas hésité, en conséquence, à renforcer leurs soutiens financiers au secteur agricole. Ils ont compris qu'aucune souveraineté forte ne pourrait se fonder hors véritable souveraineté alimentaire. Il est tout à fait consternant de constater que l'Europe s'engage sur un chemin rigoureusement inverse. Au lieu de proposer une politique à même de relancer la compétitivité des exploitations et leur capacité à investir et à se transformer, elle préfère abaisser massivement son soutien à l'agriculture. Ce désengagement sans précédent aura inévitablement des conséquences économiques désastreuses. N'oublions pas, comme nous avons eu trop tendance à le faire ces dernières années, que la PAC est avant tout une politique économique : son budget n'est pas destiné à fournir une rente aux agriculteurs, il sert essentiellement à compenser la différence entre leurs coûts de revient, qui sont fonction de standards de production les plus élevés au monde, et les prix du marché. PAC est censée permettre aux agriculteurs de dégager des marges suffisantes pour fournir l'ensemble des biens publics attendus d'eux par nos concitoyens et qui ne sont pas rémunérés par le marché, notamment au niveau environnemental. Gardons à l'esprit que sans durabilité économique il ne saurait y avoir de durabilité écologique. Sans les aides de la PAC, nombre d'exploitations agricoles françaises dégageraient un revenu négatif. Or la proposition de la Commission reviendrait, selon certaines analyses, à une diminution, en termes réels, de plus de 10 % des paiements directs et de plus de 25 % des crédits du développement rural, soit une perte d'environ 15 de la valeur totale du budget de la PAC au cours des sept prochaines années. Cette évolution se traduira par une forte détérioration du revenu final des agriculteurs, et ce tout particulièrement dans les filières les plus fragiles où le revenu des exploitants est souvent exclusivement constitué des aides de la PAC. De plus, ce tableau d'ensemble doit être complété par l'approfondissement annoncé de la convergence des paiements directs entre États membres

Comment, dans ces conditions, accepter une telle atrophie des concours publics, alors que, en 2016, près de 20 % des agriculteurs français ne pouvaient se verser de salaire et que 30 % d'entre eux touchaient moins de 350 euros par mois ? Monsieur le ministre, cette proposition de budget agricole pour la période 2021-2027 n'engage ni plus ni moins que la pérennité de certaines filières et la survie économique de nombre d'exploitations à travers notre pays. C'est donc avec une particulière gravité que nous devons aborder les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui. Une gravité qui appelle, en premier lieu, une parfaite sincérité des positions de chacun. Cela vaut pour la Commission européenne qui, par un procédé pour le moins détestable, a tenté d'avancer masquée en présentant une baisse largement sous-estimée des crédits agricoles. Ses artifices comptables jouant sur la prise en compte de l'inflation et sur les effets du Brexit n'auront toutefois pas tenu bien longtemps. Cela vaut également pour le gouvernement français. Nous avons été particulièrement troublés par les informations et les annonces du commissaire Oettinger, que nous avons reçu

ses fonctions, qui justifient et légitiment un budget substantiel pour 2020 et de conserver une politique européenne forte. Cet amendement vise donc à rappeler les objectifs de souveraineté alimentaire, de résilience et de durabilité de l'agriculture mis en avant par le Sénat dans la résolution européenne du 8 septembre 2017 sur l'avenir de la politique agricole commune à l'horizon 2020. Quel est l'avis de la commission ?

Le droit de la concurrence ne permet pas actuellement de privilégier l'approvisionnement en produits alimentaires locaux dans les procédures de marchés publics. Or, pour des raisons économiques, sociales, sanitaires et environnementales, il apparaît important d'autoriser et de favoriser le développement des circuits de proximité dans l'alimentation, notamment dans le cadre de la restauration publique. ces approvisionnements offrent une meilleure traçabilité des produits, des garanties de fraîcheur, une plus grande flexibilité limitant le gaspillage alimentaire et un faible impact carbone.

S'ils n'entrent pas dans la définition de la politique agricole commune et des règlements concernés, les circuits de proximité doivent être défendus au niveau européen par le Gouvernement. Pour ces raisons, la commission a émis un favorable

est à M. Dominique Théophile. Par leur éloignement, leur vulnérabilité au changement climatique et, pour certains, leur insularité, les régions ultrapériphériques, les RUP, sont confrontées à des obstacles qui entravent leur intégration dans le marché intérieur, rendent difficile la fourniture de produits alimentaires et agricoles essentiels et handicapent la compétitivité des filières agricoles locales. La réduction des crédits annoncée dans le projet de la Commission concernant le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2021-2027 menace les filières agricoles des RUP. Par cet amendement, il s'agit de demander le maintien d'un budget stable pour le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, communément appelé le POSEI,

l'amendement présenté par mon collègue Théophile. Nos productions doivent être protégées, compte tenu de leur vulnérabilité et des coûts induits par l'éloignement des centres d'approvisionnement et de commercialisation. Elles sont d'ailleurs qualifiées de « RUP ». Pour ce faire, une aide spécifique existe, le POSEI,

un engagement a été pris : « Nous allons poursuivre les programmes POSEI pour l'agriculture- je ne compte pas les réduire et les corriger vers le bas. »

11 millions d'euros pour les RUP françaises ! Nos économies sont fragiles, soumises à des contraintes de structure contre lesquelles on ne peut pas agir : l'éloignement, le surcoût des approvisionnements, le surcoût du fret à l'exportation,

n'ajoutons pas de l'incertitude aux incertitudes et éclaircissons définitivement le ciel de nos producteurs en stabilisant ces aides, non, que dis-je, cette compensation légitime sans laquelle nos pays seront définitivement privés de toute production endogène ! Très bien ! Je mets

à son niveau actuel. Il a été rendu public la semaine dernière à Madrid, en présence de six États : l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, la Finlande, la Grèce et la France. Je m'emploie,

Les agricultures européenne et française sont trop fragiles pour que l'on puisse accepter des coupes claires dans le budget. La PAC ne doit pas servir, cela a été dit, de variable d'ajustement du budget européen, au prétexte de la mise en oeuvre de nouvelles politiques ou du Brexit.

accroître les stocks de 4 pour 1 000 au niveau mondial contrebalancerait les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, dans l'atmosphère

L'Union européenne peut jouer en la matière un rôle important. L'INRA a d'ailleurs évalué le potentiel d'augmentation du stockage du carbone dans les sols agricoles au niveau européen à 115 millions de tonnes par an. Dès lors, si l'on rémunérait les agriculteurs qui feront l'effort d'augmenter ce stockage à hauteur de 30 euros la tonne, le coût pour la PAC tournerait autour de 3 milliards d'euros, soit 6 % du budget, avec un double bénéfice : lutter contre le changement climatique et fertiliser les sols. Ce serait un bel exemple pour le reste du monde, qui devra nourrir d'ici à quelques années 9 milliards d'habitants.

En application de l'article 73, alinéa 7, du règlement, la résolution que le Sénat vient d'adopter sera transmise au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.